La séance est ouverte. Le compte-rendu intégral de la séance de mercredi 10 mai a été publié sur le site internet y a-t-il des observations. Je n'en vois pas le procès-verbal est donc adopté. À l'ouverture de cette séance, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Roger Lise. Qui fut sénateur de la Martinique de 1977 à 1995. À présent l'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales la parole d'abord à monsieur Fabien Genêt. Merci monsieur le président, monsieur le président, Monsieur le Ministre. Chaque semaine, je rencontre les élus municipaux de mon département, de la Saône-et-Loire et je suis marquée par leurs difficultés à boucler les plans de financement de leurs investissements. Bien sûr il y a le coût de ces projets avec l'inflation et le coût des matières premières mais il y a aussi la difficulté à trouver des cofinancements et en particulier auprès des fonds européens dans un département rural comme le nôtre. Nos élus étaient habitués aux fonds Feder au fond leader et aujourd'hui ces fonds européens gérés par les régions pose aujourd'hui de grandes difficultés aux collectivités notamment rurales qui souhaite les utiliser. En effet, ces dossiers sont très complexes, il demande une ingénierie particulière dissuade bien souvent les élus à se lancer dans ces demandes dans le délai moyen de versements et de décaissements des aides et de 2 à 3 ans, ce qui était parfaitement insoutenable pour beaucoup de nos collectivités. Plusieurs exemples de terrain, témoigne que le recours à ces fonds, et bien souvent délaissés par les élus qui essaie de trouver d'autres solutions de financement de leur projet ou qui sont obligés de décaler la réalisation de ceci et il semblerait qu'il y ait d'importantes disparités régionales dans l'utilisation de ces fonds européens. Disparités qui avaient été d'ailleurs relevé par un. Un rapport d'une mission d'information sénatoriale sur la sous-utilisation chronique de ces fonds européens en France, mission conduite par notre collègue Colette Mélot c'est pourquoi Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger sur l'utilisation de ces fonds sur. La répartition de ceux-ci sur le territoire, sur leur consommation mais également sur les possibles simplifications. Des démarches pour les collectivités territoriales afin qu'elles puissent les utiliser au mieux et il me serait agréable que vous puissiez en particulier. M'indiquer les chiffres de consommation de ces crédits pour la région Bourgogne Franche-Comté qui compte. Le département de la Saône-et-Loire, je vous remercie. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur gêner. La France a bénéficié d'une enveloppe de 27 8 milliards d'euros au titre des fonds européens sur la programmation 2014 2020 et de 17 3 milliards d'euros sur la programmation 2021 2027 concernant la région Bourgogne Franche-Comté sur laquelle vous m'interrogez, ce sont 1,49 1,49 milliards d'euros qui ont été alloués à la région, au titre des différents fonds pour la période 2014 2020. La seconde période évidemment est en cours et donc que les chiffres ne sont pas définitifs. La programmation 2014 2020 a été particulière qu'elle a été marqué par plusieurs crises, en particulier celle de la Covid 19. L'Union européenne a par ailleurs lancé React You. En 2020, qui a abondé les programmes du Feder du FSE ou encore du Feader, à hauteur de 47,5 milliards d'euros pour la France, cela a représenté une enveloppe de 3,09 milliards. En 2021, et une seconde enveloppe de 822 millions d'euros en 2022, la région Bourgogne Franche-Comté a ainsi reçu d'enveloppe supplémentaire de 115 millions d'euros au titre de React You répartis sur le Feder et sur le FSE l'actuelle programmation donc 2021 2027 des fonds européens a été l'occasion. De plusieurs démarches de simplification tant au niveau européen qu'au niveau national, 80 mesures de simplification été récemment présenté par la Commission européenne au niveau français et la stabilité de la gouvernance des fonds à travers la conservation des autorités de gestion de 2014 et la réduction du nombre de programmes, de 41 à 23, contribuent aussi à cette dynamique beaucoup d'espoir donc de simplification repose aussi sur la technique des options de coûts simplifié qui facilite la justification des dépenses par les porteurs de projets et vous pouvez compter sur le gouvernement pour continuer à défendre toute mesure visant à simplifier l'instruction des dossiers. Je vous remercie. très rapidement. Je vous remercie Monsieur le Ministre de ces informations. Je regrette que vous n'ayez pas accès votre réponse sur la consommation de ces crédits. Parce que c'est là le bât qui blesse et effectivement je partage avec vous les espoirs que ces crédits puissent être mieux consommer par ce qu'il en va à la fois de l'aide aux collectivités territoriales mais également de l'image de l'Union Européenne auprès de nos concitoyens. Il y a là de défis majeurs. Merci beaucoup. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Madame. Hélène Conway Mouret. Pour sa question et pour 2 minutes. Je vous remercie monsieur le président, Monsieur le Ministre. En octobre dernier, déjà je vous interroger sur les conséquences délétères pour les relations franco-africaines de la réduction drastique des visas Louis ressortissants du Maghreb, en dépit de l'annonce de la normalisation de notre politique des visas Didier en fin d'année. Les mesures de rétorsion que la France avait adopté ont laissé des stigmates et la situation ne semble toujours pas stabilisée. Un exemple, la baisse de 30% du nombre d'apprenants à l'institut français de Tanger illustrent la lente dégradation de nos Liens d'amitié et le profond ressentiment de famille pourtant francophones et francophiles, qui préfèrent pour certaines se tourner vers d'autres pays qui leur octroie sans difficulté un VISA Schengen. Six mois se sont écoulés. C'est d'un autre pays dont je voudrais vous parler qui va servir d'exemple concret, il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Il s'agit du Cameroun ou les difficultés entourant les demandes de visas pour la France ne cesse de s'aggraver. Elle commence avec l'impossibilité d'obtenir un rendez vous puisque seuls 50 places sont proposées pour environ 500 demandes par jour afin d'apurer les retards. Le poste a sollicité des renforts. Il fait le choix de passer par un prestataire dans la gestion des prises de rendez vous dans le numéro. De téléphone dédié semble injoignable à Yaoundé des officines privées continuent à bloquer des créneaux et à les revendre à des tarifs exorbitants à des personnes qui pour des raisons professionnelles, familiales ou médicales doivent impérativement se rendent en France. Il apparaît donc que les mesures annoncées par votre ministère en décembre dernier. Non pas les effets escomptés. Tout comme les conseillers des Français de l'étranger de la circonscription je suis régulièrement saisi. Par des compatriotes dont le ou la conjointe ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour un VISA de court séjour en France. Monsieur le Ministre, je vous allez alertent régulièrement sur le besoin urgent de renforcer les équipes consulaires afin d'alléger la surcharge de travail des agents que je constate lors de chacun de mes déplacements, je voudrais vous faire une proposition ne serait-il pas envisageable de permettre à minima pour les demandes de visas de court séjour. Le dépôt du dossier par voie électronique puis de consacrer l'entretien avec un agent à l'observation des originaux et à la vérification de la conformité des pièces, je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour la réponse. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Mesdames. La sénatrice que mourir. Vous avez raison de pointer la situation d'engorgement de certains services des visas et nous la suivons avec la plus grande attention. Nous cherchons d'ailleurs sans cesse à l'améliorer ses causes sont multiples. À la hausse des demandes consécutives à la sortie de crise sanitaire, notamment pour les longs séjours s'ajoute l'exigence accrue en matière de lutte contre la fraude demandée par le ministère de l'Intérieur mais aussi l'intervention des officines que vous relevez dans certains pays d'ailleurs, le ministère se mobilisent, qu'on ne ce phénomène en communiquant auprès du public et par la mise en place d'obstacles techniques à cette captation de masse des rendez-vous par les officines. Voilà et donc la limite étant bien sûr que ces officines ne sont pas illégales. Dans les pays concernés. Enfin je ne méconnais pas les enjeux d'organisation et de fonctionnement de notre réseau consulaire. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur ont confié une mission d'expertise à Paul Hermelin assisté des corps d'inspection des deux ministères son rapport vient d'être remis et des conclusions en seront rapidement tiré à mon ministère déploie aussi des personnels temporaires pour réduire au au mieux les délais s'agit également de prioriser les publics cibles de notre politique d'affluence l'externalisation de la collecte des dossiers de demande est en place dans 46 pays, dont le Maroc et le Cameroun pour l'Automne 2023 en récupérant en amont les données biométriques en assurant que le public soit correctement informé Elle permet aussi aux agents consulaires de se concentrer sur leurs tâches régaliennes d'instruction des demandes s'agissant de la dématérialisation des procédures France VISA, l'un des 50 projets stratégiques de l'État dans le domaine des systèmes d'information vise précisément à moderniser la gestion des demandes de visas tout en renforçant sa sécurité. Ce projet doit permettre à l'usager, comme vous l'appelez de vos voeux une transmission dématérialisée du dossier cette possibilité déjà accessible pour les demandes de visas pour étude et sera progressivement étendue, enfin l'adoption prochaine de règlement européen sur la numérisation des visas permettra au traitement des demandes de courts séjours de franchir une nouvelle étape dans la dématérialisation. Je vous remercie. La. Mise au point de la représentation du gouvernement. Donc nous reprenons monsieur car dont vous avez la parole pour votre question. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre. Alors qu'une première allaite avait été lancée en octobre dernier. Quant aux dysfonctionnements de la plateforme MaPrimeRénov du constatons qu'une situation ne s'améliore toujours pas. Il y a un mois, la défenseure des droits Claire Hédon. Affirmé devant les. La commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation thermique que les difficultés d'accès à ma prime Rénov'était toujours pas résolu. Depuis. Octobre dernier, ce sont des centaines de signalements supplémentaires qui ont été reçus par d'ailleurs leur nombre à près de 1500 la plateforme MaPrimeRénov. Souffrent de graves dysfonctionnements techniques récurrents et identifiés accès dépôt de pièces impossibles sur la plateforme annonce d'inéligibilité lors de la demande de versement de l'aide alors que les travaux sont réalisés délais interminables absence encore d'information ou ou argent non versé. Ces problématiques techniques vont ralentir, voire rendre impossible. Les travaux de rénovation énergétique alors qu'il y a une urgence, une urgence car ça peut entraîner des conséquences sociales dramatiques soit ça aggrave la situation des ménages modestes. En attendant le versement de leur aide, soit c'est les plonge dans d'autres ménages d'autres ménages Et mis en place un accompagnement renforcé pour les les dossiers en difficulté les plus anciens, rien n'est fait concernant un problème de majeur de MaPrimeRénov'. Il y a une rupture des d'égalité devant le service public qui persiste avec justement l'obligation de passer par un portail Internet et le refus de mettre en place des canaux alternative au 100% numérique pour constituer les dossiers. Monsieur le Ministre, alors que les dysfonctionnements se multiplient et que les urgences sociales et climatiques se font de plus en plus pressante, comptez-vous enfin ouvrir les guichets physiques dans les espaces rend service pour rétablir l'égalité d'accès au service public de la rénovation thermique merci. À la question de monsieur, non. Avec grand plaisir. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur cardons. Vous m'interrogez sur les difficultés d'accès à l'aide financière ma prime Rénov'en matière de rénovation énergétique. Il faut rappeler que cette subvention principales aides de l'État pour accompagner les ménages en leur projet de rénovation énergétique a permis de soutenir plus de 1,5 millions d'usagers. Depuis son lancement en janvier 2020 pour répondre à ces volumes très importants tout en traitant chaque demande individuelle pour s'assurer de son éligibilité Lana mobilise des équipes dédiées pour l'instruction et le paiement des dossiers autour d'une plateforme nationale dans un contexte de forte demande et de montée en puissance du dispositif avec l'extension des publics éligibles en 2021 et les primes exceptionnelles dans le cas du plan de résilience gaz en 2022, certaines demandes ont pu c'est vrai rencontrer des difficultés à aboutir dans les à aboutir dans les délais habituels. Mais le nombre de cas est très limité. Si on le compare aux 630.000 primes engagé en 2022 par exemple l'Lana se mobilise par ailleurs très fortement pour fluidifier le parcours usagers avec la mise en place d'une équipe dédiée aux situations les plus difficiles, les dossiers en difficulté notamment ceux signalés par la défenseure des droits font l'objet d'un suivi individualisé pour résoudre au plus vite ces situations ainsi sur les quelque 500 dossiers signalés par la défenseure des droits en octobre 2022, 91 ont déjà pu être accompagnés dans leur démarche, les autres sont en cours de traitement. Lana mettent ainsi tous les moyens nécessaires en oeuvre pour assurer la qualité

d'environ 3 semaines pour obtenir le paiement lorsqu'un dossier nécessite des documents justificatifs complémentaires ou fait l'objet d'un contrôle sur place pour lutter contre la fraude. Ces délais peuvent être allongé peuvent effectivement atteint 3 mois. Il s'agit donc pas de nier les difficultés, mais de les ramener à leur juste proportion dans un dispositif dont le succès est indéniable et qui est un pilier de notre politique de rénovation énergétique. L'amélioration de la formation des usagers est aussi une priorité avec l'objectif d'accompagner l'augmentation du volume des projets de rénovation ainsi la création du service public France rénove en 2022, complété par la montée en charge progressive de mon accompagnateur et 9 en 2003 permettra de faciliter le parcours des ménages dans leur projet de rénovation. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, il vous reste 13 secondes, chers collègues. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous avez pas répondu à ma question, ma question était la suivante, est-ce que vous allez mettre en place dans les France service des accompagnateurs Hanovre pour. Aider nos concitoyens sur le le montage de dossiers, que je ne peux, je peux répondre à votre question au couple de retraités de la somme qui a dû contracter un prêt à un taux de 15%. Parce que justement il n'avait pas le versement d'aides et parce qu'il n'avait pas de nouvelles de vos services. Donc si vous voulez, je pense qu'au bout d'un moment on ne peut plus attendre, il faut agir. Si cher collègue. Nous passons à la question de mal Merzoug. Allez. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, instaurée en 2011, la taxe pluviale a été abrogée en 2015 en raison d'un coût de collecte supérieur à son rendement. permettre devait permettre de financer les installations de gestion des eaux pluviales urbaines pour l'entretien, l'exploitation le renouvellement et les extensions par la même occasion limité le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Depuis 2015, donc la gestion des eaux pluviales relèvent de la compétence des communes et des EPCI cependant aucun nouveau moyen de financement n'a été mis en place pour remplacer cette taxe. Le coût élevé de cette gestion fait que ce manque de moyens constitue un problème majeur pour des petites communes problème que confirme le budget du syndicat mixte intercommunal d'assainissement sud de la bise en Moselle. Ce sont 134.547 euros qu'ils doivent budgétés pour 2023. Or pour couvrir ses coûts. Ils ne peuvent que refacturée chaque commune. Ainsi, ce sont des factures de 45.122 euros pour la commune de AMSOW iceberg et de 13.651 euros pour Geert qui leur sont parvenues. Ce sont des communes de moins de 3000 habitants. Madame la ministre, la suppression de cette taxe entraîne des conséquences financières plus qu'importante pour les petites communes rurales. Communes qui font déjà l'objet d'autres difficultés économiques, financières, vous le savez madame la ministre, c'est pourquoi je vous demande quelles sont les bases de calcul utilisées pour déterminer le coût refacturée aux communes. Et pourquoi ce coup de gestion n'est-il pas directement intégrés dans les charges d'assainissement depuis l'abrogation de la taxe pluviale je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Dominique Faure pour sa réponse. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Herzog. Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines constituent aujourd'hui une compétence obligatoire des métropoles des communautés urbaines et des communautés d'agglomération pour les communautés de communes cette compétence est exercée à titre facultatif. Compte tenu de la faiblesse de son utilisation et sa complexité la taxe de gestion des eaux pluviales a été supprimé. Lors de l'examen de loi de finances pour 2015, le service public de gestion des eaux pluviales, ne peut être financé par une redevance. Et il est à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice en effet il n'est pas possible d'identifier la consommation de chaque usager du service de la gestion des eaux pluviales comme on peut le faire pour l'assainissement de l'eau il n'est ainsi pas possible d'établir pour le service de gestion des eaux pluviales une redevance proportionnée à l'usage du service à des abonnés dès lors qu'il s'agit d'un service rendu à l'ensemble du territoire. Par conséquent, la redevance établi pour financer le service public d'assainissement ne peut pas dans le même temps financer le service de gestion des eaux pluviales. Dès lors que la piste a été pardon expérimenter sans succès et que le service public de gestion des eaux pluviales est un service public administratif. La solution est d'en rester au financement par le budget de l'EPCI de la commune. Par ailleurs s'agissant des bases de calcul utilisées pour déterminer le coût refacturée aux communes le syndicat doit être en mesure d'isoler les dépenses Revlon relevant du seul service de gestion des eaux pluviales à ce titre l'article R-22 26 du code général des collectivités prescrit aux syndicats d'identifier l'ensemble des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines. Dans l'attente. Je me tiens à votre disposition pour rencontrer avec vous monsieur le maire de cette commune de moins de 3000 habitants pour regarder ce que l'on peut faire concrètement. Merci. Me Herzog. Il vous reste quelques secondes. Madame la ministre. Ben je retiens. Votre invitation. Donc ça sera avec plaisir que je me mettre en relation avec ces communes qui ont besoin d'être éclairé sur cette situation. Merci beaucoup. C'est à présent à monsieur Alain Dufour de poser sa question. monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette question s'adresse à Madame le la ministre chargée des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire en effet de mon département. Est traversée par 2 routes nationales. La route nationale 124 et la route nationale 21. Il s'avère que le Chef-lieu de du département. Oh, je n'ai pas relié encore à une 2 fois 2 voies ou une autoroute à la capitale régionale. Toulouse, contrairement aux autres départements. Il faut savoir que à mai 2021. Une réunion a eu lieu un protocole est intervenu à entre le l'État, le département en présence du 1er ministre qui prévoyait la achat l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale entre Auch et. Toulouse. Or à ce jour, les travaux devaient être dans d'être terminé en 2027. Ils ont effectivement commencé. En ce qui concerne la, la route nationale 21, c'est la route de. Jusqu'à, jusqu'à l'Espagne. Cette route est particulièrement accidentogène, il s'avère que rien n'a été prévu dans le cadre des plans précédents. Or, madame la ministre ma question est la suivante, est-ce que vous pensez qu'il y aura suffi dit des fonds pour prolonger la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 124 pour arriver à l'autoroute A65. Un dépeuplement. Massif et une un déclassement de cette partie de notre territoire. Par ailleurs, sur la route nationale 21, il y aurait des aménagements importants à faire, notamment en ce qui concerne le contournement de la ville d'Auch, dans le cadre de la réalisation du nouvel hôpital. voulez les quelques questions que je voulais vous poser. En espérant que vous pourrez m'apporter des réponses et de d'apporter en définitive tout apaisement à mes concitoyens hier soir qui m'interroge merci. Madame le ministre, vous répondez. à 2 fois 2 voies de la RN 124 entre Toulouse et Auch fait partie des priorités de l'État en Occitanie de premiers travaux ont pu être réalisés grâce au protocole de mai 2021 entre l'État la région Occitanie et le le département du Gers. Cet aménagement pour les ah pour l'État, vocation à être poursuivi dans le cadre de la future contractualisation du volet mobilité du contrat de plan État État-Région avec la mise à 2 fois 2 voies de la dernière section bidirectionnel entre Gimont et L'Isle-Jourdain. Une mise en service de l'infrastructure en 2027 être. Envisageable si les collectivités territoriales confirment leur intérêt pour le projet dans un contexte de crédit routier limité, vous évoquez l'hypothèse d'un aménagement à 2 fois 2 voies de la RN 124, à l'ouest d'Auch. La loi d'orientation des mobilités préconise des aménagements ponctuels plutôt que des mise à 2 fois 2 voies systématique pour les itinéraires de désenclavement l'opportunité d'un tel projet qui n'a pour l'instant fait l'objet d'aucune étude par les services de l'État reste à confirmer. Le département du Gers futur gestionnaire de l'infrastructure suite à la mise en oeuvre de la loi 3DS pourra s'il le souhaite poursuivre des études dans ce sens. Les autres aménagements que vous évoquez en particulier sur la RN 21 sont, comme vous le rappelez en discussion entre les acteurs locaux en vue de permettre au département du Gers, de disposer d'une stratégie d'aménagement partagé pour la voirie qui l'a souhaité se voir transférer je vous remercie. Très bien. Votre temps de parole mon cher collègue était entièrement consommée. La parole est à maintenant à Madame, Catherine Dumas pour sa question. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Madame la Ministre comme sénatrice de Paris Madame la Ministre je souhaite par votre intermédiaire attirer l'attention du ministre délégué en charge des transports sur les multiples nuisances occasionnées occasionnés par le dispositif de vélos taxis de type tuk-tuk à Paris une multiplicité d'infractions au code de la route est régulièrement constatés par les forces de l'ordre signalisations tricolores ne. Utilisation du portable en conduisant stationnement gênant, absence d'immatriculation de ceinture de sécurité à l'arrière, sans oublier la circulation interdite dans les couloirs de bus ou les pistes cyclables la majorité de ce type de vélos, taxis et l'ensemble des faits répréhensibles se concentre d'ailleurs dans les secteurs touristiques du centre de Paris, Trocadéro Champ-de-Mars Tour Eiffel, Louvre Tuileries. Je m'inquiète de l'explosion du nombre de véhicules tuc tuc présents dans les rues de la capitale ces derniers mois une augmentation qui d'ailleurs s'ajoute à une pratique commerciale abusive dont sont victimes de nombreux touristes français et étrangers. J'ai déjà sollicité à plusieurs reprises, les services de la préfecture de police de Paris. À ce sujet le 27 avril dernier, une opération a permis la destruction d'une trentaine d'engins illégaux mais le préfet de police de Paris m'a informé que l'action des forces de l'ordre se heurte à un vide juridique qui ne lui permettrait pas de mener une action pleinement efficace il semble notamment que des articles du code des transports requiert pour leur application un décret au Conseil d'État. Alors Madame la Ministre l'ensemble des textes qui font aujourd'hui défaut. Vont-ils enfin être publié par vos services pour permettre au préfet des actions de plus grande ampleur et arrêter ce fléau ce fléau à Madame la Ministre c'est c'est à votre parole matin. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Dumas. Je tiens tout d'abord à rappeler que le terme tuk-tuk recouvre 2 types de véhicules distinctes dans le code des transports, les véhicules motorisés à deux ou trois roues d'une part et les cycles à pédalage assisté avec assistance électrique inférieure à 0 25 kW/h d'autre part, les premiers sont régies par l'article L. 31 23 tirer 1 du code des transports et dispose d'une réglementation complète sur les obligations des entreprises qui les exploitent. Les seconds, les vélos à assistance électrique sont régies. Par l'article L. 31 23, tiré de du code des transports qui a instauré un encadrement du transport de personnes à titre onéreux. Avec de tels véhicules l'usage de véhicules relevant de ces 2 catégories et d'ores et déjà soumis au respect du code de la route dans les règles telles que le respect de la signalisation tricolore, l'interdiction de l'utilisation du portable pendant la conduite ou du stationnement gênant par exemple sont opposables à tous les usagers de la route les cycles à pédalage assisté ne sont pas autorisés à circuler ou stationner sur la voie publique en attente de clientèle. C'est une prérogative réservée aux taxis et les sanctions sont d'ores et déjà prévu dans le code des transports aux articles L. 31 24 tiré 11 et elle 31 24 tiré 12 les sanctions à la cour à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les dispositions du code de la route ou encore les dispositions générales en matière de transport de particuliers sont d'ores et déjà applicables sans texte complémentaire. Enfin, je tiens à souligner que le préfet de police et ses services sont très fortement mobilisées pour lutter contre ces pratiques irrégulières que vous mentionnez des actions de contrôle sont régulièrement réalisés et des sanctions appliquées. Je ne manquerai pas de remonter votre question personnellement à Monsieur le à Monsieur le Ministre délégué aux Transports. comme élu de Paris. Cette question me tient à coeur parce qu'il est important de trouver des solutions à ce fléau, alors que 15 à 20 millions de visiteurs vont venir à l'occasion des Jeux olympiques dans la capitale et que le monde entier aura son regard sur la capitale. Merci beaucoup. Monsieur Marc qui s'est à présent à vous. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre l'accessibilité aux services publics au statut un enjeu d'égalité et de cohésion sociale face à l'évolution de nos modes de vie et des technologies, l'organisation de nos services publics doit être repensé. Aussi, je me félicite que la mise en place du réseau France service vise à rapprocher le service public des usagers et à proposer à ceci une offre élargie de services au plus près des territoires en particulier dans les zones rurales même si c'est prévu bien évidemment aussi pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ultramarins. Car être au plus près des populations et de primordial, piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le réseau des structures labellisé France ce service se compose de près de 2400 guichets uniques de proximité regroupant plusieurs administrations sur leur site les financements d'État pour les maisons prend service vont se poursuivre à la fin de la convention les liant à la collectivité locale communes ou intercommunalités. Aussi je vous remercie de bien vouloir m'indiquer pour combien de temps ce sera le cas et à quelle hauteur. Ils vont être renouvelé. Merci, cher collègue, la parole est à la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Marc. Donc comme vous l'avez indiqué, le réseau des francs service initiée en 2019 par. Président de la République représente un nouveau modèle d'accès au service public pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen, quelle que soit l'endroit où il vit à la ville à la campagne d'accéder au service public et d'être accueillis dans un lieu unique par des personnes formées et disponible pour effectuer les démarches du quotidien depuis les premières labellisations 2020. Le gouvernement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la c'était à accompagner les collectivités pour l'implantation de nouvelles maison France Service partout sur le territoire. Nous arrivons d'ici la fin de l'année à 2750 espace France service. Et donc nous tiendrons l'engagement présidentiel. Ce dispositif a fait ses preuves. C'est pourquoi le gouvernement souhaite en assurer la pérennité. Pour cela, ce sont 12,5 millions supplémentaires qui ont pu être investis pour 2023 afin de renforcer la participation de l'État à hauteur de 5000 euros pour les France service or postal au-delà du renforcement de la participation de l'État, nous renforcerons également la qualité de l'offre de service et là les Verts pour nos usagers, vous pouvez compter sur notre totale volonté pour pérenniser ce dispositif qui a fait ses preuves. Mais pour répondre plus concrètement à votre question, il faut attendre la loi de finances 2024. Ça n'est plus qu'une question de temps Monsieur Marc. Oui, merci, madame la Ministre. Quand quelque chose ne va pas nous le disons quand quelque chose fonctionne bien et c'est le cas pour les maisons fera un service je vais encore à des collègues et tout à l'heure et qui sont présidents de comme comme qui sont maire de de petite commune de 1000 habitants, 2000 habitants, ils sont tous très heureux de ce service et cela fonctionne bien et c'est vrai qu'ils ont besoin parce que certains certains atteignent aujourd'hui la limite certains auront fini leur conventionnement à la fin de l'année et c'est pour cela que les questions ont été posées quid. Que vont devenir les agents si on n'est pas si on n'a pas la somme. Qui était cette année je crois de 35.000 euros par maison. Ce service, pour que dans le cadre du PLF bien ces sommes soit reconduites. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à madame Brigitte Lherbier. Madame le ministre, madame la secrétaire d'État auprès de la première mini chargé de l'enfance. Est venu dans le nord et changer la préfecture avec les élus et le personnel du département du Nord pour constater combien la situation des enfants. En détresse en En détresse en grand danger dans leur famille et désespérant. 270 enfants doivent être placés par ordonnance judiciaire on le rappelle régulièrement ici dans l'hémicycle en vain, faute de place dans les foyers occupés par. Les mineurs étrangers isolés. Faute de recrutement des assistantes familiales était actuellement très très difficile de recruter. Alors c'est dans ce contexte. Très douloureux pour la enfance dans le nord. Que je voulais vous parler Madame de de la protection sociale des enfants issus de la communauté rom. La la protection n'est absolument pas assurée. Victime de racisme banalisé parmi les populations les plus défavorisées d'Europe. Les Roms et plus particulièrement les mineurs ne sont pas accompagnés ni protégé par les pouvoirs publics. On estime à 15.000 le nombre de Roms sur le territoire national, dont la moitié sont des mineurs. Or ces populations extrêmement vulnérables, pour la plupart ne sont pas suivies médicalement. Ils sont en grande précarité médicale. De nombreux enfants sont contraints sous nos yeux. Mendier toute la journée dans les grandes villes et notamment à Lille, seul ou accompagné par des proches, plus ou moins douteux parfois dès le berceau. D'autres cas infiniment plus grave nous font état de proxénétisme chez les mineurs de ces populations sous les yeux de nous tous. Aussi, madame, je tenais à vous le rappeler. L'État doit à tout prix s'emparer de ce sujet. Sans une action forte. De notre part ces enfants et leurs enfants après eux resteront victime sert. De l'exclusion de la précarité mais surtout de la délinquance ne les abandonnons pas, parce que la ville n'est habilité de ses enfants nous éclate en pleine figure. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice l'herbier. Le gouvernement protège partage pleinement vos préoccupations sur la situation de ces enfants concernant les populations originaires d'Europe de l'Est qui vivent en France dans des campements et bidonvilles. Je précise que la France conformément à ses principes républicains inscrit dans la Constitution ne désigne pas une communauté sur la base de son origine. Donc je reprends concernant les populations originaires d'Europe de l'Est qui vivent en France dans des campements et bidonvilles une profonde transformation de l'action publique a été engagé dès 2018 avec une instruction du gouvernement signé par 8 ministres visant à sortir du cycle des évacuations suivi de réinstallation. L'objectif est de parvenir à une résorption définitive des lieux d'habitat informel par une action le plus tôt possible et par une approche globale intégrant prévention des risques sur les sites. Protection de l'enfance insertion sociale dont la scolarisation avec solution de relogement mais aussi sécurité publique dans un équilibre entre accès au droit et respect des lois de la République, c'est une action de très longue haleine, car elle concerne des personnes souvent déjà marginalisé dans leur pays d'origine. Elle se heurte aussi à des résistances s'expliquent en souvent par la force de l'anti-si Ghanime formes de racisme spécifique désignés comme telle dans le plan 2023 2026 de lutte contre le racisme, présenté en janvier dernier par la Première ministre. Alors des progrès sont enregistrés avec une baisse de près de 3000 personnes vivant dans ces bidonvilles et plus de 3200 enfants scolarisés grâce notamment à la création récente de 42 postes de médiateurs scolaires qui font le lien entre les familles et l'école et qui contribue ainsi à casser la spirale de la reproduction de la grande précarité. Il nous faut poursuivre bien évidemment. Merci madame la ministre et la parole est à présent et notre collègue Jean-Baptiste blanc.

Il a été doté de 2 milliards d'euros de crédits les destinées à financer des projets présentés par les collectivités regroupement qui vont dans le sens de la transition écologique avait 14 sous-thèmes qui vont de la prévention des inondations à la renaturation des villes et villages. Hé bien encore ou bien encore le le recyclage des friches. Les élus étaient très enthousiastes sont toujours pour déposer des dossiers, mais depuis quelques temps, quelques critiques quelques doutes se font entendre. Il y a un besoin de plus de transparence et de simplification de toute évidence, ce fonds a été répartis entre les territoires en fonction de critères démographiques et de leurs besoins propres, mais la répartition entre les territoires. Et la répartition au sein d'un même territoire ne sont pas toujours connues. Or ce fonds Vert sera un succès ne sera un succès que si il bénéficie équitablement à tous les territoires qu'ils soient ruraux urbains périurbains littoraux montagne et bien sûr à toutes les catégories de collectivités. En outre, les préfets de région sont chargées en toute liberté d'attribuer ce fonds Vert ou pas aux collectivités selon des critères qu'ils décident eux- mêmes alors certes avec les, les préfets de département parfois. Mais c'est une critique récurrente qu'on entend chez les élus locaux, au même titre que les enveloppes de dotation d'équipement des territoires ruraux la DETR, ainsi que la déciles il commanderait que les réponses et notamment les réponses négatives soit. Car il serait fâcheux que ce fonds Vert viennent en réalité pallier les insuffisances. Des dotations DETR décile et qui ne sont en vérité qu'une DETR déciles repeinte en Vert. Il est et les besoins sont immenses pour faire face aux défis climatiques. Il était donc impératif de reconduire ce ce fonds et c'est ce qui vient d'annoncer la Première ministre ou le 3 avril, mai 2. Faudrait faudrait-il pas aller plus loin, c'est la 2ème. Question qui se pose, cette somme ne devrait-elle pas être globalisé. Pluriannuel et non fléchés projet par projet, tant les besoins sont immenses. Contrairement à la première mouture ou les maires de France avait n'avait pas c'était associés en amont. Le gouvernement a annoncé le lancement d'une concertation avec les associations d'élus. L'occasion sans du dos de réfléchir au besoin de transparence, simplification réclamée par les élus comme par exemple répondre avec les soucis de logiciels. Ce qui remonte souvent qui a pas qui apparemment pose problème et peut être. Prioriser les besoins en réduisant le nombre de thèmes. Il faut donc je souhaitais vous interroger là-dessus sur toutes ces pistes d'amélioration que l'on pourrait envisager ensemble. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre c'est à vous de répondre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur blanc. Donc le ministre Christophe Béchu a voulu un dispositif souple transparent et des. Il est souple et transparent, car nous avons fait des cahiers d'un complément d'accompagnement éducatif est partagé entre les porteurs de projets et les instructeurs chargés d'analyser de hiérarchiser les demandes il est déconcentrée pour que le Fonds Vert s'appuie sur le dialogue territorial. Au total ce ce sont 4 milliards d'euros qui sont engagés par l'État. 2 milliards aussi de la DETR, et de là d'ici les 2 milliards anti-du Fonds Vert pour accompagner les collectivités dans la transition écologique à travers le Fonds Vert et les dotations d'investissement. L'impact écologique et recherché sur tout le territoire 1417 demandes sont situés en zone de revitalisation rurale 578 ans quartiers prioritaires les 2 tiers sont portés dans des communes de moins de de 10.000 habitants, la mobilisation des élus s'observe dans tous les départements ainsi que dans les collectivités d'outre-mer en ce qui concerne l'accompagnement des porteurs de projets. L'outil démarches simplifiées un guide disponible via la plateforme et territoires avec de multiples ressources d'information enfin de répondre aux attentes des porteurs de projets. L'administration du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a été chargé de mener les concertations nécessaires pour tenir compte de l'expérience de ces premiers mois des échanges réguliers ont par ailleurs lieu entre le gouvernement et les préfets afin de perfectionner ce dispositif. Les associations d'élus ont été consultés. Dès la création du fonds 20 et demain je les recevrai à nouveau aux côtés de Christophe Béchu pour échanger notamment sur la pérennisation du fonds Vert en 2024 comme annoncé par la Première ministre le 3 avril, l'accélération de la transition écologique se fera dans les territoires avec les collectivités locales grâce à l'engagement de tous leurs élus pour les soutenir, ils peuvent compter sur le fond Vert cependant j'entends les propositions et les améliorations que vous portez. Je me tiens avec Christophe Béchu à votre disposition pour en parler et travailler. Améliorer le dispositif. Si Madame la Ministre. La parole est à présent madame Sylvie Robert. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Le 24 avril dernier, la maire de Rennes et les présidents des différentes associations de commerçants de cette ville ont adressé à la Première ministre un courrier relatant les grandes difficultés commerciales, financières et assurantiel traversée par ces commerçants et artisans situé en centre-ville. En effet, ils ont subi d'importants dégâts liés notamment à la violence d'éléments extérieurs à la mobilisation contre la réforme des retraites. Ici il les bien essentiel de rappeler que ces dégradations y compris que le contre le mobilier urbain pourtant bien public et ses troubles alors de public ne doivent en aucun cas à mal d'être amalgamé avec toutes les manifestations qui ont été organisées par les syndicats et qui se sont très bien déroulées en 2016, Rennes a fait aussi face à une situation aussi singulière qui appelle une réponse singulière pour aider et accompagner ces commerçants et artisans doublement victime, victime d'importants préjudices matériels et de lourdes pertes d'exploitation. La baisse du chiffre d'affaires des commerçants du centre-ville est estimé à 41 millions d'euros pour le tu remets trimestres 2023 victimes aussi d'un défaut de couverts. Assuranciel qui se manifeste notamment par la résiliation unilatérale de leur contrat par les assureurs et par l'insertion d'une clause ainsi durant une période probatoire de 2 ans son cynisme. Dans le cas des contrats nouvellement proposé. En 2016 le gouvernement avait rapidement réagi en remboursant les franchises et en débloquant une aide exceptionnelle pour compenser les pertes d'exploitation et préserver l'activité économique et l'emploi. Madame la Ministre, êtes-vous prêt à aller dans le même sens et à soutenir les commerçants et artisans de Rennes en mettant en place un fonds de compensation. Êtes-vous également prête avec vos collègues de l'économie et des finances, à faire évoluer la loi afin que les assureurs ne puissent plus rompre unilatéralement les contrats dès lors que les dégradations sur le fait de casseurs isolés. Vous savez, les commerçants et les artisans subissent ainsi une double peine. C'est une affaire de justice, mais aussi de sauvegarde ne nos centre-ville. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la ministre. C'est à vous. Merci monsieur le président, mesdames, vous allez, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice. Robert la loi et la jurisprudence reconnaissent déjà au commerçant rennais comme à toute personne victime de dégradations liées à la violence de casseurs. La possibilité d'obtenir de plein droit la prise en charge par l'État des préjudices qui n'aurait pas été indemnisées indemnisées par leurs assureurs. Ils peuvent en effet utiliser de régimes distincts de responsabilité sans faute de l'État. D'une part l'article L 211 tirer 10 du code de la sécurité intérieure ouvrant droit à indemnisation pour les victimes de dommages intervenus lors d'attroupements ou de rassemblements d'autre part le régime jurisprudentielle de responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que la victime établie qu'elle a subi un préjudice grave et spécial qui ne saurait être regardée comme une charge lui incombant normalement résultant notamment de la fermeture de commerce pour prévenir leur saccage. À cet égard depuis 2019 l'État à indemniser à hauteur de 14,5 millions d'euros, dont plus de 6,7 millions en 2022. Les victimes de dommages causés lors des manifestations et notamment les commerçants et dans la plupart des cas de façon amiable démontrant ainsi que ces régimes de responsabilités nous paraissent suffisants pour assurer l'indemnisation de toutes les victimes. Je vous remercie. Monsieur disons c'est à vous. En particulier dans le département de la Moselle dans ce territoire l'isolement des agriculteurs permettait effectivement à large spectre de délit gasoil siphonnés Vol de fioul de métaux tracteurs dérobé puis abandonné dégradé acte de vandalisme. Voitures brûlées ou encore Vol d'animaux. Détail d'importance, ces actes délictueux surtout ce sont souvent le fait de jeunes délinquants ceux interpellés récemment dans le cas de la commune de blouson ville toujours en Moselle ont entre 14 et 16 ans. Et que dire des nombreux vols de GPS, outil précieux à plus d'un titre. Ce matériel de géolocalisation et d'auto-guidage par satellite qui permet aux agriculteurs de gagner en temps en précision et par là même en productivité coûte en moyenne 10.000 euros. Conséquence, les GPS, c'est cool. Très bien et très vite au marché noir certains d'. Roubaix en Moselle se rallume à New York. Mais alors que médias régionaux. Et nationaux confondus. Dénonce cette situation et donne la parole aux victimes comme à ce céréaliers éleveurs mosellans de trop bornes toujours en Moselle, le phénomène gagne en importance. Aussi, madame la ministre, entendez-vous mettre en place une politique de sécurité spécifiques à nos territoires ruraux avec davantage d'effectifs de gendarmerie spécialisé dans cette catégorie de vol. Je vous remercie. Si cher collègue, la parole est à l'ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Mison. S'inscrivant dans une logique. Partenariat avec le monde agricole, la gendarmerie nationale décline au niveau national et dans chaque territoire une politique de sécurité ambitieuse en matière de lutte contre les atteintes aux exploitations agricoles, elle comprend plusieurs volets, de la prévention à la répression en passant par l'accompagnement des victimes. Localement, comme à la compagnie de boulets Moselle les exploitants agricoles peuvent bénéficier de l'accompagnement des correspondants sûreté présents au sein de chaque brigade de gendarmerie pour disposer de conseils de sécurisation à l'échelon départemental, la gendarmerie propose gracieusement l'expertise de ses référents sûreté en matière de sécurisation des exploitations agricoles et d'accompagnement à la mise en place de dispositifs de vidéoprotection. La gendarmerie informe également sur les phénomènes d'appropriation et diffuse des bonnes pratiques lors des réunions d'information au profit des représentants de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et des Jeunes Agriculteurs. De plus, la gendarmerie s'investit dans le traitement judiciaire des atteintes aux exploitations agricoles, les enquêtes diligentées par les les unités de police judiciaire de la gendarmerie permettent de mettre un coup d'arrêt aux activités de groupes criminels. Au niveau central, un suivi particulier de ces atteintes est effectuée par le Service central de renseignement criminel de la gendarmerie et permet d'en dresser des analyses opérationnelles qui sont relayées vers les échelons territoriaux de commandement de la gendarmerie. La direction générale de la gendarmerie nationale adapte la réponse de la gendarmerie aux besoins de sécurité exprimés par la profession actuellement dans un souci constant d'amélioration de la prise en charge des victimes. La gendarmerie développe un dispositif de prise de plainte en mobilité, c'est-à-dire aux 10.000 au domicile du du plaignant, permettant ainsi aux agriculteurs victimes de déposer plainte sans avoir à se déplacer en brigade de gendarmerie je me permets de rajouter que les 200 brigades. Nouvelle et qui vont être annoncés sur les mois de juin et juillet permettront en renfort générale qui s'appliquera plus particulièrement ruralité auprès des agriculteurs. Monsieur maison ne disposer de plus de 20 secondes pour votre réponse. Merci monsieur le président. Je vous remercie. Madame la Ministre je vous remercie pour votre réponse. Elle est sur un plan intellectuel. Très satisfaisante mais sans casser que les réponses qui satisfont l'esprit ne règle pas forcément les problèmes, c'est en tout cas ce qu'on constate. Sur le terrain je j'ai évoqué la question du matériel agricole. J'aurais pu évoquer celle du BTP ou le constat est similaire. Et je pense, je pense que vous ne ferait pas l'économie d'un renforcement encore supplémentaire pour venir à bout ce drame qui déchire et qui se fait tant souffrir, nous. Nos campagnes. Merci. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dite loi MAPTAM du 27 janvier 2014, précise la compétence des EPCI en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Des inondations pardon, la fameuse Gemapi en France métropolitaine linéaire recensés de digues à entretenir et de 6000 kilomètres. Ces dernières peuvent se trouver à cheval sur plusieurs EPCI aussi, la loi prévoit elle un délai complémentaire pour le transfert de cette compétence dans ce cadre un certain nombre de communes actuellement gestionnaire rencontrent des difficultés à faire reconnaître l'utilité des systèmes d'endiguement à leurs EPCI réputé à terme compétents. Dans le Sauternais en Gironde les rives de la Garonne sont sauvegardés par un système d'endiguement construit en 1855. Depuis 150 ans ces Terres protégés ont été habité cultivé et bien sûr. C'est C'est tout particulièrement le cas des systèmes d'endiguement de tout laine prennent et prennent Jacques Barsac à cheval sur 2 communautés de communes convergence Garonne et Sud-Gironde. Depuis 2014, ces systèmes d'endiguement abrite de stations d'épuration, dont celle qui traite les effluents vinicoles de tout le Sauterne et un stade municipal, une portion de la route départementale 11 13 et une trentaine d'habitations. Ces digues ont fait l'objet constant d'effort financier considérable de la part des collectivités et de l'État pour être entretenu améliorer et même reconstruite suite à la crue de 2021. Pourtant l'une des 2 intercommunalité s'est d'ores et déjà prononcé le 4 avril dernier à bulletins secrets contre la prise de compétence de ces digues la 2ème CDC doit voter le 31 mai prochain et l'inquiétude des maires concernés et grande. Que se passera-t-il si elle refuse également cette compétence ou qu'elle l'accepte sans couvrir toutefois la totalité des travaux ce qui serait normal. C'est pourquoi madame la Ministre je trouve souhaiterais savoir ce que le gouvernement peut faire pour débloquer cette situation et éviter a minima une gabegie des deniers publics, au pire une catastrophe humaine. Je vous remercie. Merci cher présidente pour votre exactitude Madame la Ministre vous ferez aussi bien. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice de Lattre la compétence de gestion des inondations et de prévention des inondations. La Gemapi a été confiée par la loi MAPTAM aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette compétence obligatoire doit permettre d'assurer la bonne gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Les inondations ne connaissent pas les frontières administratives. C'est pourquoi de nombreux systèmes d'endiguement sont à cheval sur plusieurs communes, la gouvernance de la compétence Gemapi doivent donc pouvoir s'adapter pour garantir à l'échelle appropriée la cohérence de l'action publique en matière de prévention des inondations. La loi MAPTAM a prévu des outils destinés à faciliter la gouvernance de la Gemapi dans le respect du principe de libre administration des collectivités pour gérer chaque système d'endiguement l'échelle la plus pertinente pour les fêtes. L'efficacité de la protection d'un territoire la loi donne la possibilité aux EPCI à fiscalité propre de transférer la compétence ou même seulement de la déléguée un syndicat mixte spécialisée de type. Établissement public territorial de bassin ou de type établissement public de gestion et d'aménagement de l'eau, c'est en particulier le cas pour un système d'endiguement qui dépasserait le territoire du seuls EPCI à fiscalité propre. Par ailleurs, une digue non reprise dans un système d'endiguement doit être neutralisée pour éviter tout accident lors d'une crue par le dialogue qu'ils assurent avec les collectivités, les préfets de département veillent à ce que les choix de gouvernance de celle-ci n'aient pas de conséquences négatives pour la pérennisation des endiguement utile à nos concitoyens en 2023 le gouvernement spécifiquement défini des mesures du Fonds Vert. Parmi les 14 critères. Pour accompagner les territoires qui pourraient rencontrer des difficultés financières ces aides vise comme vous le soulignez à ce que des systèmes d'endiguement utiles à la protection contre les inondations ne soit pas abandonnée. Je vous remercie. Merci de me rappeler au bonheur de cette à Pierre-Jean Verzeletti de de prendre la parole avec mes plates excuses.

c'est des. Cette décision signifie que les bailleurs devront respecter une réglementation stricte de sécurité incendie. Celles applicables aux établissements recevant du public, ce qui va remettre en cause le développement de l'habitat actuel L'habitat inclusif, lancée en 2017 par la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel constitue une forme d'habitat adapté pour beaucoup de personnes âgées. Ou dépendantes ou en situation de handicap. C'est un intermédiaire entre le logement ordinaire et l'accueil en établissement. En pratique, il s'agit de plusieurs logements indépendants adapté est caractérisée par la volonté de ses habitants de vivre ensemble. Ces derniers signent un bail, ce qui en fait des locataires, comme les autres. Le gouvernement a récemment réaffirmé sa volonté politique de développer ce modèle domiciliaires sur l'ensemble du territoire. Cependant, l'avis du Conseil d'État interroge la future dynamique de déploiement de ses habitants inclusif. Cette mise en conformité, va concerner les habitats inclusif regroupant plus de six personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap. Or pour fonctionner de façon optimale ces habitants ont besoin de plus de six personnes afin de faciliter la mutualisation de ressources et permettent le recrutement d'une personne présente 24h sur 24. Cette Cette décision va également avoir des conséquences sur le développement de l'habitat inclusif de façon totalement contradictoire avec la réforme souhaitée par le gouvernement. En effet, les bailleurs sociaux vont se montrer beaucoup plus frileux et examiné plus sérieusement le risque de loger loger des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap. Enfin cette décision remet en cause le développement de l'habitat inclusif en ce qu'ils constituaient une étape structurant de la transformation de l'offre au bénéfice de l'inclusion des personnes en situation de handicap. De nombreux projets s'étaient déployés en accord avec les aspirations de vie des personnes concernées et représenter un espoir pour beaucoup d'entre eux. Aussi, j'appelle le gouvernement à une mise en cohérence des réglementations en matière d'habitat inclusif afin de répondre aux enjeux de ce modèle et d'assurer aux occupants des habitants inclusif un soutien indéfectible. Merci. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Vert laine. La juridiction administrative a considéré que la concentration en un lieu unique de personnes dans l'aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie est nécessairement diminuer et que cette aptitude. Et constitutif des paramètres à retenir pour l'appréciation des mesures en vue d'assurer la sécurité des personnes contre l'incendie. En vertu de l'article L 143 tiré 3 du code de la construction et de l'habitation, les espaces destinés à loger des personnes handicapées constitué donc un établissement destiné à recevoir du public au sens de la réglementation de sécurité quand contre l'incendie. Le fait que les personnes handicapées concernés soient titulaires d'un contrat de location et ne soit pas admise dans un établissement médico-social et que l'immeuble ne comporte pas de lieux collectifs de vie ne faisait pas obstacle à cette qualification de RP. En conséquence, mes services ont engagé sous un format interministériel des travaux pour faire évoluer la réglementation applicable à ce type de logement. Des échanges entre nos services et ceux du ministère en charge de la construction et du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont en cours et devraient aboutir. Ah une soumission juridique complète les différents acteurs du secteur sont également associés à cette démarche. Une telle réglementation doit concilier le développement légitime de l'habitat inclusif sur l'ensemble du territoire national avec la nécessaire préservation de la sécurité de tous les occupants de ces logements ainsi que des services de secours appelés à intervenir en cas de sinistre. Le cadre juridique devra prévoir des prescriptions spécifiques pour garantir un niveau de sécurité contre les risques d'incendie adapté à ce type d'habitations et de public. C'est pour ces raisons. Monsieur le sénateur que le gouvernement envisage de compléter le corpus juridique applicable en matière de protection incendie des logements et tout et tout particulièrement des bâtiments accueillants de l'habitat inclusif. Je vous remercie. Très bien malin la miss. Merci beaucoup et la parole à présent hé bien à Stéphane Demilly. Merci, monsieur le Président, bonjour, madame la Ministre. L'article 1612 2 du code général des collectivités locales, stipule que le budget primitif des collectivités doit être adopté avant le 15 avril, sauf années bien sûr de renouvellement ou un délai supplémentaire de 15 jours est accordé. Les articles 2612 1 et suivants, liste les documents que les services de l'État doivent transmettre aux décideurs concernés avant l'adoption du budget afin notamment bien sûr de contribuer à la sincérité du scénario budgétaire. Or Madame la Ministre nous constatons que le délai entre la réception de ces informations et la Deadline du vote officiel se réduit comme peau de chagrin. Mon collègue Jean hein grève vous avez d'ailleurs déjà alerté sur ce sujet l'année dernière, sans détailler le calendrier de notification de toutes les dotations prenons simplement l'exemple le plus emblématique, celui de la DGF depuis plusieurs années, son montant communiqué aux conseils municipaux. La première semaine d'avril, ce qui ne laisse plus qu'une semaine pour le cas échéant réunir la commission des finances et planifier la séance de conseil municipal. Sachant que le délai de convocation du conseil et de 3 jours francs pour une commune de moins de 3500 habitants et de 5 jours pour les autres, ce n'est plus une peau de chagrin. Madame la Ministre c'est une vraie seringue. Vous me répondrez. Peut-être qu'il est possible de repousser la date de vote en cas de réception tardive je cite des informations indispensables à l'établissement du budget. Ce qui nous rappelle ce qui nous rapproche pardon du milieu de l'année civile, ce qui vous en conviendrez n'est pas acceptable. Cette situation est particulièrement problématique pour nos communes, vous le comprenez Madame le Ministre des aménagements sont-ils prévus afin que les collectivités puissent recevoir leurs informations budgétaires et ainsi voter leur budget annuel dans un délai un peu plus raisonnables. madame la ministre, votre réponse. Et pourtant, monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Demilly. Les collectivités territoriales et de leurs groupements doivent voter leur budget, vous l'avez dit avant le 15 avril de l'année, cette date intervient 15 jours après transmission par l'état des éléments utiles à la préparation de ce budget dans la liste est fixé par décret. Si ces éléments utiles sont transmis après le 31 mars, vous l'avez dit, la loi dispose que la date limite de vote des taux est décalé afin de laisser un délai d'examen d'au moins 15 jours aux collectivités territoriales pour voter leur budget, je vous le rappelle, vous l'avez dit mais c'est pas ma réponse est un élément de ma réponse, je tiens à souligner le délai contraint. Parce que quand on est de. C'est intéressant de connaître les contraintes de l'autre partie. Et donc le délai contraint dont disposent les services de l'État pour effectuer la répartition de la DGF du fait d'une part, de la disponibilité tardive de certaines données et d'autre part de la complexité de la répartition de près de 27 milliards d'euros à l'euro à l'euro près selon des règles complexes reposant sur un grand nombre de critères physiques, financiers et sociaux et je l'ai vécu cette année cette complexité parce que j'avais moi-même insisté pour que l'on avance dès cette année, cette date d'information des DGF à nos collectivités chaque année tous les efforts sont mis en oeuvre. Par les services de la direction générale des collectivités territoriales pour publier le plus tôt possible les résultats de la répartition de la DGF en 2020 malgré les très fortes perturbations engendrées par la crise sanitaire, la publication est intervenu le 6 avril en 2021. La publication a eu lieu le 2 avril. Cette année pour la première fois la mise en ligne est intervenue. Le 31 mars. Et comme je me suis engagé auprès de votre collègue sénateur, j'ai demandé au service pour l'année 2024 de raccourcir le délai de la répartition et de prévoir sa publication. Une semaine plus tôt, soit le 24 mars, ils s'y sont dans petit à petit. Je pense que nous allons vers plutôt un mois que 15 jours on sera trois semaines en 2024. Je vous remercie. il vous reste 14 secondes pour vous en réjouir. Monsieur le sénateur Madame Filleul, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre dans mon département du Nord, la commune de Saint Saulve vit une situation financière particulièrement difficile, liées au calcul de sa dotation globale de fonctionnement et peine à sortir la tête de l'eau. Monsieur Yves Dussart sommaire le dénonce depuis plusieurs années auprès de l'État et de ses représentants, sans que rien ne change jamais. Je serai car je ne suis pas la première parlementaire à me saisir de ce sujet, d'autres collègues députés ou sénateurs sont déjà intervenus en hémicycle à chaque question toujours les mêmes réponses. Le gouvernement reconnaît que la situation est anormale, mais rien n'est fait par avance, je vous prie, madame la Ministre, de ne pas gâcher le précieux temps de réponse que vous avez pour nous dire encore qu'il s'agit du poids de l'histoire concernant le calcul de la DGF ou de ne pas rentrer dans des explications techniques connues de tous, vous les connaissez, les élus le savent déjà, nous le savons tous, déjà de fait, c'est une question d'égalité de traitement d'autant que le président de la République a déjà débloqué des fonds exceptionnel de par le passé, je pense à celui reçu par exemple par la ville de Marseille. Les élus légitimement ne comprennent pas ce 2 poids 2 mesures, je vous demande donc une réponse concrète à la question suivante, allez-vous oui ou non apporter une aide immédiate à la commune de Saint Saulve en quelque sorte son du. Le maire de la commune, croyez-le bien, Madame fort et le 1er à écouter votre réponse je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la ministre vous avez la parole. Merci monsieur le président. Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Sophie, la commune de Saint Saulve perçoit une DGF par habitant inférieur à la moyenne des communes de la même strate de population, c'est-à-dire 40 euros. Quatre par habitant en 2023 contre une moyenne de la strate de 168,6 euros. Le niveau relativement faible de la DGF de Saint Saulve est lié à son attribution et vous l'avez indiqué au titre de la dotation forfaitaire qui s'établit à 8 euros. Huit par habitant en 2023 contre une moyenne nationale de 93,3 euros. Cette inégalité de DGF provient pour partie et vous l'avez indiqué. De la consolidation de composantes historiques figée dans la dotation forfaitaire à la suite des réformes successives si les modes de calcul ont ainsi été simplifiées autour de l'évolution de la population communale des écarts historique de dotations entre communes sont maintenus et explique cette inégalité intrinsèque, elle ne nous satisfait pas. Depuis 2017, le poids de la dotation forfaitaire qui cristallise les plus fortes inégalités dans la DGF des communes a été réduit au profit des dotations de péréquation. Or les dotations de péréquation sont répartis en fonction de critères objectifs de ressources et de charges indépendant des choix de gestion des communes et qui font l'unanimité. C'est d'ailleurs l'évolution de ces dotations de péréquation qui permet la DGF de la commune de Saint Saulve de progresser de 4,4% en 2023. Je vous rejoint dans le constat de la nécessité d'une réforme de la dotation forfaitaire des communes, nous y travaillons. Une telle réforme produire et tout. Toutefois, des variations à la hausse ou à la baisse de la dotation forfaitaire de nombreuses communes de ce fait, j'ai demandé qu'une large. Concertation soit menée dans le cadre de l'agenda territorial avant de l'engager. Nous nous y sommes attelés avec Christophe Béchu et avec la DGCL je vous remercie. Madame Filleul, il vous reste. Un moment de réponse. Oui, je vous remercie beaucoup Monsieur le Président, je vous remercie également Madame la Ministre de vos éléments de réponse. Néanmoins vous comprendrez qu'il ne me satisfont pas car il n'y a pas de réponse concrète précise dans l'urgence pour la commune de Saint-. Qui est vraiment en attente et par conséquent, moi je ce que je suis obligé de constater, c'est que vous ne vous engagez pas à venir au secours de cette commune qui est en grande difficulté. Oui, oui. Madame même le le gouvernement prend la parole. Je vous remercie. Et contrairement à ce que vous venez de dire, je m'engage bien évidemment à venir au secours de cette commune si elle est en difficulté. La question de la DGF est un sujet je suis à votre disposition, comme je l'ai proposé pour recevoir monsieur le maire avec la DGCL et nous travaillerons sur la façon dont nous pouvons accompagner cette commune si. Elle est en difficulté, je vous remercie. Très bien. La parole est à présent madame Cathy pour ce. Merci monsieur le président, madame la ministre, je ne peux commencer mon propos sans avoir évidemment une pensée pour le maire de. Saint-Brévin-les-Pins. Victime d'une violence extrême qui l'a conduit à démissionner de sa fonction de nombreux maires de nombreux élus de la République m'interpelle dans mon département le Pas-de-Calais puisqu'ils sont eux aussi parfois victimes et cible d'individus de groupuscules qui les insultes ou les agressent physiquement Madame la Ministre je pense qu'il faut prendre des mesures plus énergiques pour ne pas laisser en souffrance, ses élus, madame la Ministre, en octobre 2022 lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2023, le gouvernement a décidé de venir en aide aux collectivités les plus fragilisées pour qu'elle puisse faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires en instaurant le filet de sécurité. À ce jour nous sommes interpellés par plusieurs maires qui risque de devoir rembourser la ont perçu. Trouvez-vous ça juste. Quelles mesures comptez-vous prendre pour ne pas pénaliser les efforts consentis par ces collectivités. Première question pour vous pouvez-vous m'indiquer Madame la Ministre combien de communes sont impactées dans le Pas-de-Calais. Par ailleurs, la dotation exceptionnelle de DGF pour 2023 n'est pas accompagnée par une revalorisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale DSU qui augmentent moins vite que l'inflation 1,7 compte 6% cela induit une perte de capacités financières pour les villes les plus pauvres, enfin vous le savez, les maires et notamment les maires ruraux souffrent du manque de moyens humains ils sont souvent amenés à à traiter l'ensemble des dossiers et des problématiques avec le leur seul secrétaire de mairie aujourd'hui plus que jamais la question d'un guichet unique se pose celui-ci faciliterait l'accès aux aides aux subventions et surtout aux interlocuteurs adaptés aux problématiques qui les touchent en effet ce n'est pas faire offense aux maires et aux secrétaire de mairie que de dire qu'il ne l'est plus, de plus en plus compliqué de s'y retrouver entre les compétences des uns les prérogatives des autres. Qu'avez-vous effectivement prévu à ce sujet au sujet évidemment du guichet unique. Je vous remercie, madame la Ministre. Madame la Ministre c'est à vous de prendre la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice a pour. Beaucoup beaucoup de questions. Je crains de pas pouvoir répondre dans le temps imparti à toute n'quelques mots pour soutenir les collectivités territoriales face aux effets de l'inflation et les aider à investir dans la transition écologique, un ensemble de mesures ont été mises en oeuvre en loi de finances pour 2023, parmi lesquels une hausse de la DGF pour la première fois depuis 13 ans, vous le savez, 320 millions d'euros en 2023 d'augmentation. L'État considérablement renforcé son soutien à l'investissement dans les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure les dotations de soutien à l'investissement local sont maintenues à 2023 à l'heure au niveau historique de 2 milliards d'euros le fond d'accélération de la transition écologique des territoires a été créé et doté de 2 milliards d'euros supplémentaires. Il sera reconduit en 2023, le gouvernement a déployé plusieurs mesures de soutien face à la hausse des dépenses d'énergies payés par les collectivités territoriales à travers plusieurs dispositifs. Je ne vais pas les les énumérer en détail mais le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité le filet de sécurité. Et là vous me dites c'était. Dans le PLFR 2023 on a voté 430 millions d'euros et on a versé des acomptes aujourd'hui vous me dites, trouvez-vous normal qu'on reprenne les acomptes dans cette loi de finances assorti à ses 430.000 millions d'euros. Il y avait des critères. Or nous avons payé rapidement. C'est ça compte mais en indiquant qu'il fallait s'assurer que les critères étaient bien respectées et donc oui je trouve normal que quand des acomptes ont été versés à tort bien il puisse être repris. Donc tous ces sujets, c'est, c'est évidemment un peu de, de bon sens sur le sujet de. La revalorisation globalement du métier. Des secrétaires de mairie, on travaille avec Stanislas Guerini. À une revalorisation globale de ce métier par un renforcement de l'offre de formation par une promotion spécifique des agents dans le cadre de leur parcours professionnel et par une reconnaissance de leur contribution essentielle aux élus. On travaille sur comment on va pouvoir mettre en place ces formations et à quelle échéance au pouvoir, proposer aux maires des promotions de jeunes et nouvelle secrétaire de mairie. Au-delà de la revalorisation de leur statut et de leur rémunération. Je vous remercie. Merci madame la ministre. La parole est à présent madame Amel Gacquerre. Qui clôt une longue série de sénateur du haut de France. Monsieur le Président Madame la Ministre. Le 9 mars dernier à Béthune Nadège. Une mère de famille de 48 ans a été victime de féminicides tué à son domicile par son ancien compagnon sous les yeux de sa fille âgée de 12 ans. Il y a près d'un an. Toujours dans le Béthunois 2 enfants âgés de 4 et 7 ans, était retrouvé mort dans une voiture incendiée par leur père. Ce dernier n'avait pas supporté la séparation avec son ex-conjointe. Ces deux drames récents dans le Pas-de-Calais parmi de nombreux autres malheureusement ont un point commun, l'auteur des crimes était connu des services de police et des et de gendarmerie. Force est de constater qu'a aujourd'hui les dispositifs de protection des victimes et la réponse pénale sont insuffisants. À Béthune, la femme tuée par son ex-compagnon avait porté plainte pour menaces de mort 8 mois avant son assassinat. Selon le collectif Féminicides, 31 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année 2023. La plupart des auteurs avait fait l'objet de dépôt de plainte, voire même de condamnations trop souvent les délais allongés entre le dépôt d'une plainte pour violences et la réponse du parquet place la victime dans une situation de danger durant laquelle nombre de conjoints ou ex-conjoints violents passent à l'acte. Pour sécuriser la situation des femmes qui portent plainte. Il serait notamment impératif de fixer un délai maximal entre le dépôt de plainte et la réponse du parquet qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'un classement sans suite, il faut le reconnaître. L'État a sensiblement augmenté les moyens alloués à la lutte contre les violences conjugales. Or, le nombre de violences conjugales augmente toujours et les inégalités territoriales demeure la région Hauts de France est la plus touchée par les féminicides. Il est essentiel d'adapter la lutte aux réalités locales de territorialiser les politiques et d'augmenter les moyens mobilisés Madame la Ministre quels outils et moyens supplémentaires comptez-vous mettre en oeuvre rapidement pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, notamment dans les territoires les plus touchés par ce fléau ici, Les Hauts de France que prévoyez-vous pour renforcer la protection des victimes et améliorer la réponse pénale afin d'éviter de nouveaux drames. Je vous remercie. La parole vous revient. Madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice gars depuis 2017. Le gouvernement a lancé une mobilisation générale de l'État en lien avec les associations et les collectivités pour lutter contre le fléau des violences intrafamiliales. Le gouvernement a lancé en mars le déploiement du Pack nouveau départ qui a vocation à apporter une réponse coordonnée rapide et individualisé aux besoins des victimes de violences conjugales en vue de les aider à quitter leur conjoint violent. Ces victimes seront ainsi mieux détecter grâce à un réseau d'acteurs de première ligne sensibilisés et formés. Il permettra une priorisation de l'accès aux aides et dispositifs de droit commun comme un. Une logique. Coupe-file il comprendra notamment la possibilité d'une aide financière d'urgence ce Pack nouveau départ sera élargie à la France entière d'ici fin 2025. Par ailleurs, le 8 mars, le gouvernement a présenté le plan toutes et tous égaux. Ce plan comporte plusieurs mesures pour lutter contre le fléau des violences intrafamiliales dans les territoires, notamment le déploiement de pôles spécialisés dans chaque juridiction, le renforcement de la formation des magistrats. Et de l'ensemble des acteurs de première ligne en matière de lutte contre les violences intrafamiliales donc déploiement de pôles spécialisés, renforcement de la formation des magistrats en cas de danger grave et imminent en pour les victimes une ordonnance de protection immédiate pourrait être délivré sous 24h. Le fichier carrément de protection des victimes de violences intrafamiliales sera enrichi progressivement des données relatives à la victime pour mieux la protéger. Enfin, chaque département sera dotée d'une structure médico-sociale de prise en charge globale des femmes victimes de tout type de violence, adossé à un centre hospitalier afin de généraliser le recueil de plainte le gouvernement consacrent des moyens budgétaires et humains sans précédent à la lutte contre les violences conjugales. Le budget du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes a été multiplié par 2 ces 5 dernières années. Pour autant, il nous faut poursuivre, il nous faut accélérer et il nous faut progresser ensemble, merci, je vous remercie. Merci, madame la Ministre, la parole est à présent à Madame, Cristina Pucher pour sa question. Merci monsieur le président, mes chers collègues. Madame la Ministre. Le gouvernement a lancé début mars auprès des fédérations professionnelles concernées une consultation pour modifier l'arrêté qui fixe les conditions d'obtention du Label basse consommation je fais référence ici au dispositif lié à ma prime Rénov'. Est ainsi envisagée, l'exclusion je cite des chaudières alimentées majoritairement par des combustibles combustibles fossiles. Nous ne sommes pas naïfs, il s'agit là d'une première mesure allant dans le sens du projet de règlement de la Commission européenne, qui souhaite interdire dès 2002 toutes les chaudières, y compris compatible avec des biocombustibles alors même que les parlementaires européens sont parvenus à un compromis pour les autoriser. Or les parlementaires français vont devoir se saisir de la stratégie française sur l'énergie et le climat avec 2 échéances majeures en 2023 et 2024, ces orientations sont donc vous en conviendrez éminemment questionnable le gouvernement sans procéder à des orientations énergétiques stratégiques par voie réglementaire en amont du législateur. Ensuite Madame la Ministre sur sur cette question épineuse sur laquelle le gouvernement a été plusieurs fois interrogé, j'ai lu vos arguments. Vos, vos chiffres, vos promesses de concertation mais j'aimerais une fois pour toutes, que vous nous expliquez sur quelles études précises, vous êtes fondé pour envisager d'exclure toute un vecteur énergétique de chauffage. Qui remplira pourtant des critères très intéressant de performances, quels sont les résultats de l'étude d'impact économique que vous avez bien évidemment mener pour envisager une telle mesure d'envergure. Compte tenu des lourdes conséquences financières pour les ménages français. Il serait dommage qu'on s'aperçoive a posteriori que tout cela repose sur des projections dogmatique et incomplète comme d'autres décisions énergétiques passer. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Flucher. Il y a à ce jour pas d'interdiction d'installation de chaudière gaz dans les logements existants. Depuis le début de l'année 2022, la réglementation environnementale R. 20 20. Impose le recours à une part importante d'énergies décarbonnées pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les logements neufs. S'agissant du biogaz, énergie décarboné qui n'est pas utilisé seulement dans le secteur des bâtiments son développement doit être encouragée. Je rappelle néanmoins les ordres de grandeur jeu nous avons consommé 480 TWh de gaz en 2021 et nous avons actuellement une capacité d'injection dans le réseau de seulement 10 TWh de biogaz. Avec un gisement globale de biomasse qui restera limitée est fortement sollicité par ailleurs. Les tarifs d'achats du biogaz injecté dans les réseaux seront bientôt revaloriser et accompagné de plusieurs mesures de simplification et de flexibilisation le dispositif des certificats de production de biométhane introduit par la loi climat et résilience de 2021 obligera progressivement les fournisseurs à augmenter la part de biométhane incorporé. Réduire notre consommation globale de gaz n'est donc pas incompatibles avec un développement fort du biogaz au service des secteurs et pour le cas où les alternatives au gaz sont limités. Nous devons faire les deux. Afin de sortir au plus vite des énergies fossiles. Nous devons décarboner notre économie et nous devons renforcer notre souveraineté énergétique concernant une éventuelle interdiction progressive de la vente de chaudière gaz neuf une telle décision ne pourrait s'envisager qu'après une concertation large et documenté, avec toutes les parties prenantes et dimensionné précisément tenant compte de l'ensemble des enjeux techniques et économiques associés comme vous l'avez indiqué afin de ne laisser aucun ménage dans l'impasse. Et de donner suffisamment de visibilité à tous les professionnels, je vous remercie. Très bien. Il vous reste quelques secondes pour compléter votre intervention madame. Merci Madame le Ministre bon vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question mais moi j'ai envie de vous dire qu'il faut maintenant tirer la leçon de ceux qui passe et ce qui, de ce qui s'est passé l'hiver dernier. Soyez pragmatique le mixte énergétique est toujours plus prudent. La parole est à présent hein. Madame Agnès Canayer. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre pendant près de 50 ans. L'administration française et, mais tellement la Normandie qu'elle en avait créé de mais depuis 2015 à Normandie réunifiée au bénéfice de sa rationalité de sa performance pourtant ce rapprochement naturel demeure inaboutie. En effet, l'organisation de la justice en Normandie et tout sauf normande. Elle est tantôt nordique tantôt bretonne ainsi l'unité opérationnelle de Rouen est rattaché au budget opérationnel de programme Bob Grand Nord géré par la cour d'appel de Douai. Quant à celle de Caen elle dépend du bop Grand-Ouest relevant de la cour d'appel de Rennes. Cette organisation subordonne la cour d'appel de Rouen à 4. Cour d'appel, selon les thématiques entraînant de graves conséquences sur le pilotage de la justice en Normandie cette situation amenuise l'efficacité judiciaire. Voir l'entrave cette situation illustre parfaitement les conclusions du rapport des états généraux de la justice qui pointé la discordance entre la carte administrative et judiciaire au niveau régional, la création d'un BOP Normand est donc indispensable pour assurer l'efficience de l'action de la justice au niveau régional, tout en étant en cohérence avec le schéma territorial de toutes les autres administrations de l'État. Les acteurs Normand demande donc de la cohérence territoriale aussi, je souhaiterais connaître quelles sont les intentions du gouvernement sur ce sujet. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Canayer. Alors comme vous le savez le gouvernement, et tout particulièrement le garde des Sceaux. Sommes très attachés à la proximité de l'institution judiciaire avec les territoires. Le garde des Sceaux connaît également à la fois votre engagement pour votre territoire mais également pour la justice de notre pays. Cette question d'organisation budgétaire et comptable revêt une importance toute particulière à l'heure où il s'apprête à présenter la loi de programmation pour la justice.

La question que vous soulevez donc en lien Direct avec la transformation majeure que le garde des Sceaux porte pour la justice. L'une des clés du succès bien celle de la réorganisation des services administratifs déconcentrée. Des services judiciaires. C'est la raison pour laquelle le garde des Sceaux a demandé à l'administration de mettre en place une grande opération de déconcentration au 1er janvier 2024 aujourd'hui. Nous sommes encore en train d'envisager toutes les hypothèses pour bâtir un projet cohérent. Vous comprendrez que nous ne pouvons donner une réponse ferme sur une cour d'appel alors que nous souhaitons penser une solution plus globale. Toutefois, le garde des Sceaux garde en mémoire votre proposition particulièrement bien étayé et nous vous suggérons il vous suggère de pouvoir vous en discutez prochainement à la Chancellerie, afin d'avancer sur des propositions concrètes, je vous remercie. mais. Évidemment sur le sujet de la justice. Nous connaissons particulièrement bien ses intentions mais je tenais ce matin a attiré particulièrement là aussi. Son attention sur l'enjeu pour la Normandie de cette réorganisation dont on ne connaît pas exactement les contours. Merci, cher collègue, la parole est à présent hein monsieur Max Brisson pour sa question. Merci Monsieur président Madame la Ministre face aux sévères épisodes de sécheresse de 2022. L'état de calamité agricole a été reconnu dans les plaines Atlantique. Oui, le gouvernement a pris la mesure de la gravité de la situation en division entend un assouplissement des critères d'éligibilité dont un abaissement de 13 11 % du taux de perte du produit sur le produit brut et depuis le 16 janvier, les paysans basque et béarnais peuvent faire leur déclaration pour toucher l'indemnité compensatoire qui leur revient toutefois près de 33% des demandes déposées sur l'ensemble du département ont été rejetées, soit un éleveur sur 3 exclues du dispositif. Et pour cause. Celui-ci n'est pas adapté aux spécificités des exploitations d'élevage du département en effet les fermes ayant une surface moyenne d'environ 30 hectares surfaces relativement faible en comparaison des moyennes nationales mais elle supporte grâce à la transhumance en montagne des cheptels conséquent pour leur permettre de dégager un revenu cette singularité qui permet de classer le département. Sur le podium des installations de jeunes agriculteurs est toutefois difficilement pris en compte dans les différentes mesures d'aides conjoncturelles mise en en place les remontées de terrain indique que le seuil de 11% de perte de produit brut est trop exclure aussi Madame la Ministre pour répondre au désarroi des éleveurs, le gouvernement est-t-il enclin. À proposer de nouveaux critères des Libye Judith et aux aides accepteraient-ils au moins de fixer un nouveau seuil de perte à 8%. Conformément à la motion formulée par la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Si cher collègue Madame la Ministre, vous avez la parole. de sécheresse au travers pour le régime des calamités agricoles une accélération exceptionnelle de la procédure, plus de quatre mois gagnés au profit des éleveurs les plus affectées. Deuxièmement la décision exceptionnelle de relever le taux d'indemnisation de 28% à 35% s'agissant du département des Pyrénées-Atlantiques, le CNG R à du 9 décembre a émis un avis favorable pour la reconnaissance du département en calamités agricoles pour les pertes subies suite à la sécheresse sur fourrage le CNG du 15 mars 2023 a aussi émis un avis favorable concernant les pertes de fonds sur plan de cultures pérennes sur l'ensemble du de de votre département. J'ai conscience néanmoins que ni l'accélération du calendrier ni le relèvement exceptionnel du taux d'indemnisation ne bénéficie aux agriculteurs ils ne sont pas éligible aux calamités notamment ceux qui n'atteignent pas le seuil de 11% de perte globale. Il convient de rappeler que ce seuil a déjà fait l'objet d'un abaissement à titre exceptionnel dans le cadre de la sécheresse. 2022. Le gouvernement est donc conscient du fait que le département des Pyrénées-Atlantiques n'a pas été concerné par les sécheresses ces années passées, que le dispositif des calamités agricoles sur fourrage complexe à déployer n'est pas un outil habituel dans le département. Aussi. Marc Fesneau a demandé au service de la DDT avec l'appui des des équipes du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire de réaliser un travail de vérification approfondie des paramètres de cette calamité. Un travail d'analyse des dossiers inéligible et de vérification d'erreur de déclaration de saisie a été menée. Monsieur le sénateur, ce critère n'existe plus dans le nouveau système d'assurance-récolte en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Je vous remercie. Sauf que face à la situation est la suivante, un tiers des dossiers sont actuellement rejetées. Les éleveurs du département. La hausse actuellement, un véritable cri de détresse. Ils l'ont d'ailleurs dit au ministre Marcello ce qu'il est venu dans le département certaines exploitations sont aujourd'hui en danger alors qu'on était dans un territoire où les installations se produisait actuellement nous nous sommes en train de remettre en cause. Avec ces critères qui ne répondent pas à la réalité du département des DPD authentique. Un territoire qui avait de, de belles installations, il ne l'économie de montagne de transhumance qui était partout en performante. Donc je demande à nouveau gouvernement de regarder de près la situation des éleveurs de la montagne pyrénéenne. Merci, cher collègue, la parole est à présent aux questeur Jean-Pierre Sueur. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre je souhaite appeler votre attention sur la situation de l'Agence française anticorruption, comme vous le savez, cette agence créée par la loi du 9 décembre 2016 devait répondre notamment aux critiques de l'OCDE qui pointé je cite la faible réactivité des autorités françaises et la faiblesse des moyens affectés aux enquêtes dans la lutte contre la corruption. Or depuis juillet 2022 les 6 personnalités qui composent la commission des sanctions qui peut être saisie par l'Agence ont cessé leurs fonctions et le et leurs successeurs n'ont pas encore été nommé à ce jour, à ma connaissance. Ensuite le magistrat qui dirigeait l'Agence française anticorruption vient de terminer son mandat et la direction et donc vacante enfin une circulaire dédié au traitement des atteintes à la probité qui l'a annoncé en septembre 2022 qui devait être adressée début 2023 se fait également attendre pour toutes ces raisons je vous demande Madame la Ministre quelles décisions vont être prises afin de donner à cette agence dont le rôle est essentiel. Les moyens d'assumer sa mission. Merci cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur sueur. L'Agence française anticorruption, l'AFA, un rôle essentiel qui est pleinement reconnu et encouragé par le gouvernement français. Dans son rapport de 2021, l'OCDE souligné que la France a entrepris des réformes de première importance pour lutter efficacement contre la corruption, la fac 36 agents à sa création 2017 elle en dénombre 50 depuis décembre 2022, 5 créations d'emplois supplémentaires ont été arbitré sur la trajectoire 2023 2024 afin de multiplier les contrôles liés à la Coupe du monde de rugby 2023 et aux JO 2024 afin de renforcer les contrôles des sociétés publiques locales des entreprises étrangères opérant en France ainsi que les contrôles de suite sur les acteurs publics et sur les entreprises. La dotation globale de la fin pour ses dépenses d'expertise et maintenu un haut niveau, à savoir 350.000 euros annuels pour les années 2023 à 2027. À cette somme s'ajoutent les avances de frais d'expertise des convention judiciaire d'intérêt public qui peuvent représenter jusqu'à 2 à 3 millions d'euros par an. Le décret portant nomination de membres de la commission des sanctions a été publié le 17 avril 2023 et la nomination d'un nouveau directeur de l'agence est en cours. Le gouvernement est particulièrement soucieux de préserver des moyens alloués à louer à la fin un au niveau et de les faire évoluer en lien avec les nécessités inhérentes à la poursuite de ses missions par ailleurs une circulaire portant sur les relations entre l'autorité judiciaire et les juridictions financières sera très prochainement diffusé afin d'améliorer la détection de ces infractions et les moyens permettant de favoriser des enquêtes efficaces et une réponse pénale dynamique des travaux interministériels importants sont actuellement menées sous la coordination de la fin. Pour l'élaboration d'un nouveau plan pluriannuel de lutte contre la corruption pour la période 2023 2025. Il sera au au niveau des standards internationaux les plus exigeants. Vous pouvez compter sur nous, monsieur le sénateur, je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Sueur, vous avez la parole. Monsieur le Président. De vos déclarations. Madame la Ministre je j'espère que les six personnes composant cette commission des sanctions fonte fonte être effectivement nommé puisque le texte a fait vous dit est paru et que le directeur qui est en cours de nomination depuis déjà un certain temps finira par être nommé. Je rappelle que l'ancien directeur, a déclaré devant l'Assemblée nationale, une commission de l'Assemblée nationale que les capacités d'action et les personnels sont nettement inférieurs à ce qui était prévu au moment de de la loi 53. Effectif. Il en est, il était question de 70 voyez-vous, il faut que cela augmente et, vu l'importance du sujet, c'est absolument nécessaire. Merci cher collègue. Et merci à la ministre. Qui nous quitte et la parole est à Gilbert Roger. Pour sa question. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est une question que j'ai déposée en octobre dernier donc. La réponse. A tardé à venir jusqu'à nous. À la suite de révélations de la presse, les Français comme le Parlement ont appris la tentative de la DGFIP de faire évoluer le fichier des comptes bancaires et assimilés Ficoba. En 2021 pour y inclure toutes les informations bancaires, des citoyens français. Ce processus s'est fait dans une opacité totale telle que ni le parlement ni la Commission nationale informatique et libertés non n'avait été averti de ces démarches pourtant garante des libertés publiques, nombreux sont nos concitoyens qui se questionnent dont certains m'ont interpellé sur la tentative de Bercy de s'arroger autant autant de données personnelles sans l'accord de la représentation nationale. Aussi, merci de bien vouloir expliquer sur cette réforme qui dispose d'aucune base légale à ce jour je crois tout en détaillant la vision de Bercy. Quant à l'utilisation des informations bancaires des Français dans un futur proche. Merci cher collègue. Monsieur le ministre vous avez la parole. Merci Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, l'article. 16 49 A du code général des impôts fait obligation aux organismes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières de déclarer à l'administration fiscale, l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature, ainsi que la location de coffre-fort. Les données collectées sont répertoriés dans le fichier des comptes bancaires Ficoba détenu par la DGFIP ce fichier et consultés par les services de la DGFIP en charge du contrôle fiscal et du recouvrement ainsi que par les organismes dûment autorisé par le législateur à des fins notamment de lutte contre la fraude. Le fichier des comptes bancaires et assimilés, créé en 1971. Informatisé en 1982 et mise à jour en 2002 Ficoba 2 recense donc les comptes de toute nature ouverts sur le territoire national fournit aux organismes légalement habilité dans le cadre de l'exercice de leur mission, des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société cette application est aujourd'hui obsolète, tant sur le plan fonctionnel que technique, elle n'est pas en capacité de prendre en compte les évolutions du secteur bancaire et doit répondre à un accroissement des sollicitations. Dans ce contexte, la refonte de Ficoba est essentiel pour la DGFIP et les nombreux partenaires et acteurs en charge de la lutte contre les différents types de fraude et elle vise plus largement améliorer le recouvrement des créances publiques des études de modernisation technique et fonctionnelle ont donc été engagées, c'est le projet Ficoba trois sur la période 2022 1023 pour lesquels un financement a été obtenu dans le cadre du FTA. 2020. Le fond de transformation de l'action publique dans le cadre de ses travaux des réflexions interne à l'administration été conduite sur l'intégration ou non dans le fichier des données relatives au sol des comptes bancaires à une date donnée. Il s'agit d'une réflexion logique car disposer du solde des comptes n'est pas en soi une nouveauté conceptuelle. En effet le fichier Fico qui recense les assurances vie permet de connaître le solde de ces dernières. De même, l'administration fiscale dispose des soldes des comptes bancaires détenus à l'étranger par des résidents fiscaux français grâce aux données de l'échange automatique d'informations internationales. Une telle évolution du fichier Ficoba ne serait, en tout état de cause possible qu'après avis de la CNIL et intervention du législateur. sénateur en en septembre prochain. Mais comme il va y avoir une loi de finances. J'encourage le gouvernement actuel a déposé devant la représentation nationale. Des projets qui fasse que ce ne soit pas une réflexion technique mais bien une approbation du législateur, il ne faut pas marcher sur nos plates-bandes, merci. Merci de votre vigilance. Cher collègue, la parole est à présent hein. Gilbert Luc vinasse pour sa question. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Depuis le 1er janvier 2023, en application de la loi tous les centres de formalités des entreprises ont été regroupés sur un seul site, le guichet unique. Cela représente un défi colossal à la charge de l'INPI pour avoir rencontré la chambre des métiers de l'artisanat de mon territoire, la réalité sur le terrain est difficile depuis la mise en oeuvre de cette simplification de nombreux dysfonctionnements sont apparus les dans le désarroi des milliers d'entrepreneurs, mais aussi le réseau consulaire. Ce qui a eu pour conséquence le mécontentement le stress des mandataires des clients et des collaborateurs consulaire. Si les chambres des métiers ont perdu le rôle de service public dans la gestion de centres de former des formalités. Elle le conserve quant à la validation des déclarations prêtées par le guichet il Or il a été constaté des erreurs d'orientation d'entreprises vers les registres du commerce ou de l'art qui l'Urssaf au lieu d'être orienté vers la chambre les chambres des métiers. Cela a un impact financier pour les CM1 puisque les entreprises non inscrite à la section artisanale du répertoire national ne seront pas soumises à la taxe pour les frais de la chance. Par ailleurs la qualification professionnelle n'est pas vérifié ce qui peut porter préjudice aux consommateurs comment comptez-vous sécuriser ces aspects dans les évolutions de la plateforme unique et quand pourra-t-on compter sur un guichet unique pleinement opérationnel. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur devinettes, permettez-moi de vous apporter la réponse de mon collègue. Jean-Noël Barrot, en particulier sur l'instauration du guichet unique pour les formalités d'entreprises qui constituent à la fois où vous l'avez dit, monsieur le sénateur, un projet technique d'extrême d'extrême grande ampleur et une redéfinition en profondeur du rôle de l'ensemble des acteurs de l'écosystème des formalités après plus de 40 ans de fonctionnement des centres de formalités des entreprises, les fameux CFE ces 2 facteurs expliquent une grande partie je crois monsieur le sénateur, et il faut le dire. Des retards que le projet a connu à son démarrage et que le gouvernement s'est engagé à résorber. Ouvert en janvier dernier. Conformément à la loi pacte le guichet unique a permis aux entreprises effectivement de réaliser plus de. 845.000. Formalités depuis cette date, il prend d'ores et déjà en charge la totalité des formalités de création et ce dernier également. prend le cas des cessations dans quelques jours les tests se poursuivent actuellement pour les formalités de modifications qui ouvriront progressivement d'ici juin. Enfin une nouvelle version simplifiée et je sais que vous y tenez monsieur le sénateur du dépôt des comptes est disponible à la fin avril dans cette transformation. Les chambres des métiers et de l'artisanat qui ont un rôle absolument essentiel dans l'accompagnement des entreprises sur nos différents territoires aujourd'hui conserve un rôle extrêmement déterminant et il leur appartient en effet de vérifier le caractère artisanale de l'activité déclarée par l'entreprise c'est également elle qui doivent contrôler la qualification professionnelle. Enfin, s'agissant de l'orientation des dossiers vers les organismes en charge des validations dont le les CMA si elle se repose exclusivement sur les informations fournies par les entreprises concernant concernant leurs activités au moyen des classifications évidemment des activités et conjointement avec les chambres. Monsieur le sénateur, malgré les difficultés inhérentes à un projet d'une aussi grande ampleur que le guichet unique. Provoque d'une certaine manière, soyez rassurés sur la pleine mobilisation du gouvernement pour corriger les défauts constatés et permettre une mise en place pleine et effective le plus rapidement possible parce que c'est l'engagement que les équipes en particulier à Bercy en prise je vous remercie. Merci madame le Ministre, chers collègues, vous avez la parole. Et. Madame la Ministre veuillez m'excuser, j'avais pas vu le changement de ministre. Je vous remercie de votre réponse, simplement une remarque pour avoir avec la délégation aux entreprises du Sénat a visité ligne pays. On a écouté les explications, je pense que dans la construction de ce guichet unique. Si les chambres consulaires n'avait pas été considéré uniquement comme des acteurs, mais comme des actes des partenaires à part entière. Les choses se déroulerait beaucoup mieux. Si cher collègue, la parole est à présent à monsieur Olivier et nous pour ces questions. le cafard. Alors les causes sont nombreuses. Il y a la violence et la démission du maire de Saint-Brévin et est hautement symbolique. Les maires, les élus locaux veulent bien être à portée d'engueulade, mais pas à porter de de coups victime de de violence et l'État doit agir. Une autre cause c'est la production des normes des normes très nombreux et et Lausanne est évidemment un exemple et puis il y a la question de l'insécurité financière avec parfois une une dépendance les maires et les élus locaux veulent d'une décentralisation de projets, ils ne veulent pas une décentralisation d'exécution. Ils veulent pouvoir conduire des des des projets, ils ne veulent pas des, des agents de l'État, mais bien au contraire, ils veulent de l'autonomie fiscale et et de la lisibilité financière et c'est bien la la la la la question est donc, concernant la lisibilité financière. Ce qui se passe sur l'automatisation du faux de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impact des choix opérés par le gouvernement sur le budget des communes et hautement symbolique. En effet, l'État a décidé d'exclure du FCTVA un certain nombre de dépenses, parmi lesquels les 2 comptes d'immobilisation de m'111 terrains et 212 agencement et aménagement du terrain et cette exclusion entraîne une perte de 350.000 euros pour un certain nombre de communes et notamment la ville de Lambersart, car les dépenses sont liées à la rénovation de de terrains de sport en gazon synthétique courant 2000, Vel trois qui ne serait donc pas reprises en compte et donc je me fait part de l'inquiétude du maire de Lambersart pour ses investissements et j'appelle une réponse claire sur les dispositifs, 211 et 212. Parce que c'est un exemple très très illustratif de l'insécurité financière dont sont victimes les maires et les élus locaux. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, et nous vous avez rappelé. Les actes de violence que subissent les maires en particulier depuis le début du mandat. Depuis le début du mandat, monsieur, le monsieur le sénateur, et vous le savez, c'est presque. 1500 maires qui ont démissionné, qui ont démissionné alors qu'ils ont cette charge de faire vivre leur commune et ils se sont présentés devant devant les électeurs. Il se trouve que que on ne peut pas commencer cette réponse sans rappeler le soutien au maire de Saint-Brévin qui est de mon territoire de Loire-Atlantique et qui a vu, d'une certaine manière le pire voir son propre domicile. Incendiés et des insultes et des menaces en présence de ses enfants et je crois que personne, personne n'a accepté, ni de violence ni d'intimidation, ni qu'on soit maire qu'on soit sénateur qu'on soit député conçoit Miss qu'on est d'une certaine manière en charge une part hé bien un petit bout de notre République et de notre démocratie et monsieur le maire vous l'avez rappelé, les difficultés elles sont de divers ordres et en particulier. elle elle porte sur l'automatisation du FCTVA de manière très technique, puisque la question dans le fond est particulièrement technique. Au-delà des propos sur le ras-le-bol ou la difficulté et le vague à l'âme d'une certaine manière que peuvent avoir légitimement un certain nombre de maires quand ils subissent des violences sur leur territoire. Il se trouve que le périmètre des comptes des plans. Ne permet pas de faire coïncider exactement l'assiette automatisée et l'assiette réglementaire précédent la réforme certains comptes d'agencement et d'aménagement des terrains n'ont pas été retenus dans l'assiette automatisée car il comporte des dépenses hors taxe par nature in éligibles au FCTVA. Toutefois, Monsieur le Maire. Les dépenses réalisées par les collectivités. Dans ce cadre d'aménagement d'un terrain de sport sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du FCTVA ainsi les achats d'équipements sportifs ou urbains qu'il soit a fixé au sol ou non sont inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA et il en va de même de l'achat de machines d'entretien du terrain ou encore du matériel d'éclairage de dépenses. Monsieur le sénateur, et je vois que le temps file. Ne le permettent plus simplement le coût supplémentaire pour l'État et au-delà. En réalité, avec 7 automatiquement. Cette automatisation. Ce que je vous propose, monsieur le sénateur, puisque votre question est technique et précise c'est vous apporter par écrit aujourd'hui la réponse plus complète qui m'a été transmise parce que ça pourra apporter une réponse aux maires je crois que c'est bien l'essentiel. Je vous remercie. et notamment de la ministre de la Culture sur la situation de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie située à Darnétal dans mon département. Les INSA sont au coeur des enjeux de Patrimoine et de la cité, notamment au regard de la loi du 7 juillet, dite loi elle cap qui a contribué à réhabiliter le rôle et la place de l'architecture dans la cité et non sans une ambition conjointe avec le Patrimoine par ailleurs face au défi climatique et écologique d'aménagement aussi équilibré du territoire et d'urbanisme auquel l'ensemble de la société confrontée ainsi que de collectivités territoriales, ces écoles sont amenées à jouer un rôle non seulement en matière de formation initiale mais également continue dans une logique de réflexion et d'adéquation et d'adaptation permanente depuis plusieurs semaines, mais de même plusieurs mois l'Ensam rencontre de graves problèmes structurels, résultat d'un manque d'investissement dans la formation, l'accompagnement pédagogique et les locaux de l'école. Cela a eu pour conséquence une grève suite à une initiative conjointe entre les enseignants et les étudiants courant février. Les services du ministère ont reçu une délégation de l'Ensam courant mars, sans que soit véritablement actées, un nouveau rendez-vous concernant les futurs moyens accordés à l'école, notamment dans le cadre du prochain projet de loi de finances et ce malgré les nombreux efforts menés par la direction. S'agissant des finances et le personnel enseignant sur la transformation des formations, notamment en matière environnementale, en août l'argent public investi par étudiant moyen pour les Elsa est significativement inférieur à celui du reste de l'enseignement supérieur donc l'école de Normandie faisant de plus partie de la fourchette basse dans les moyens et ETP alloués aux INSA donc dans une logique d'équité avec les autres branches de l'enseignement supérieur face aussi à l'importance du rôle les ça pour l'avenir. Je vous demande et je demande à madame la mise à culture si elle entend allouer des moyens à la hauteur des enjeux à l'occasion du prochain projet de loi de finances voir dans le cas du 1er, projet de loi de finances rectificative de 2023. Je vous remercie pour votre réponse. merci ma chère collègue Madame le Ministre c'est boots à vous la parole. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Morin-Desailly. On connaît votre engagement particulier. Pour accompagner la situation spécifique de l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie puisque. Votre vos alertes ont été récurrentes madame là. Sénatrice et ça m'a été rappelé par le cabinet et par la ministre de la culture, donc je voulais le le rappeler ici, il se trouve que plus que jamais, nous avons besoin. D'accompagner un certain nombre. Hé bien d'établissements qui ont vocation aussi à apporter un certain nombre de réponses pour la transition écologique est le grand défi de notre siècle. La ministre de la Culture a fait c'est vrai une priorité, celui du budget 2023, je crois, en témoigne une augmentation inédite de 20% des crédits qui leur ont été consacrés. Il vient s'ajouter 57 millions pour le plan de relance de la rénovation des bâtiments. Au total les Elsa bénéficie d'un investissement de plus de 75 millions d'euros programmée d'ici 2025. Cependant, madame la sénatrice, quand j'entends votre question votre question elle pose en particulier sur l'INSA de Normandie et ben les ça en général et donc pour apporter une réponse franche et directe. Ma collègue Rima Abdul-Malak a rencontrer personnellement, les représentants des étudiants, les directeurs et les différents présidents Denza mais plus spécifiquement. La question qui se pose puisque les rencontres, date des dernières semaines c'est une large concertation qui. A notamment permis d'annoncer une aide immédiate de 3 millions d'euros plus spécifiquement. À la vie étudiante et enfin le soutien en faveur de la recherche sera accru les rémunérations des enseignants. De recherche et des doctorants dès la rentrée seront alignés sur leurs homologues universitaire au-delà de ça, madame la sénatrice et pour répondre au fond de votre question. La ministre m'a rappelé son attachement.

et réactualiser la stratégie élaborée en 2015 qui date maintenant et de l'inscrire dans les défis de notre temps aujourd'hui et je vous assure. Madame la sénatrice que je m'engage à demander à ce que la ministre vous tienne au courant. Étape après étape de ces concertations vu votre mobilisation je vous remercie. Merci, madame la Ministre de la parole est à madame Céline Brulin pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre le filet de sécurité qui doit permettre aux collectivités de faire face à l'explosion des coûts de l'énergie se traduit par des versements d'acomptes aux communes potentiellement bénéficiaires certaines on ne l'ont d'ailleurs pas demandé de crainte de devoir rembourser car c'est en effet à l'établissement du compte administratif que les collectivités connaissent avec certitude l'évolution de leur épargne brute qui doit avoir diminué de 25% pour bénéficier du filet de sécurité 2022. Les premières régularisations tombe et des communes. À l'image d'Harfleur ou de Maromme en Seine-Maritime doivent rembourser, parfois des centaines de milliers d'euros, ce qui est évidemment en péril leur équilibre budgétaire c'est injuste car ce sont leurs efforts de gestion qui conduisent précisément à une moindre diminution de leur épargne brute c'est aussi contre-productif car cela impacte les investissements par exemple des rénovations thermiques qui permettrait de diminuer durablement les coûts de l'énergie dans d'autres cas comme celui de la ville de le contrôle de légalité, pointe l'insuffisance de ressources propres de la commune au regard des coûts énergétiques mais c'est bien là le problème avec des fluctuations qui rendent difficile l'élaboration des Budgets il faut repousser la régularisation. Le ministre des Comptes publics a donné quelques signes en ce sens, je crois qu'il convient de garantir aux communes concernées qu'aucun remboursement ne leur sera demandé avant au minimum d'avoir examiné leur situation de 2023. Il faut aussi améliorer le dispositif, nous avons réussi à abaisser à 15% le critère de perte d'autofinancement pour 2023 mais le décret a été rejeté par le comité des finances locales. Parce qu'il conduisait à exclure beaucoup trop de collectivités quand et dans quel sens. Ce décret sera-t-il retravailler republié je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice brûle hein. Permettez-moi de vous apporter une réponse plutôt lu ce qui est assez rare dans ma bouche, ce que je j'apprécie pas spécialement l'exercice. Mais la question est, est particulièrement technique et donc je voudrais apporter une réponse quand même assez assez exhaustive. Effectivement, le gouvernement est pleinement conscient de cette inflation sur la situation financière des collectivités et donc agi. En lien avec le Parlement bien sûr la mise en place du c'est du filet de sécurité contre les conséquences de l'inflation figurant à l'article 14 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022. Je crois en est l'illustration. Ce dispositif vise évidemment compenser un certain nombre de hausse des dépenses en 2022 et permet d'apporter un soutien financier immédiat cependant le décret. Que vous citez, celui du 13 octobre, 2022 ans, précise le fonctionnement et un décrit les modalités de calcul de calcul et le versement des dotations octroyées à ce titre pour accompagner les collectivités les plus en difficulté. Le mécanisme d'acompte que vous connaissez allant de 30 à 50% des dotations prévues, a été mis en place à leur demande les collectivités pouvait solliciter jusqu'au 15 novembre dernier un acompte à condition qu'elles anticipent. À la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25% sur le le le fondement d'une estimation de leur situation financière. Il a toutefois été indiqué que les collectivités bénéficiaires pourraient être amenés à à rembourser l'acompte en 2023. Si au vu de l'exécution budgétaire 2022 le montant définitif de la dotation calculée est inférieur à celui de l'acompte versé en 2022 à ce stade les travaux. Et les dotations en définitive n'ont pas encore été totalement calculé et les services du ministère n'ont formulé aucune demande de remboursement d'acompte. L'article 113 de de la loi. Du 30 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 a reconduit un filet de sécurité sur les dépenses supporters 2023 en élargissant le Champ des bénéficiaires, il vise plus spécifiquement à compenser les effets de hausse des dépenses ah d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et les. Dispositions du décret prévoit un certain nombre de réponses, les mesures de soutien prévu par la loi de finances. Seront présentes, madame la sénatrice, comme pour monsieur le sénateur, je vous propose vous vous compléter la réponse extrêmement techniques extrêmement longue par écrit pour apporter un certain nombre de réponses évidemment aux maires concernés. Je vous remercie. Un homme brûle hein. Il vous reste quelques secondes pour moi si Monsieur le. Président, vous avez vu en lisant cette réponse la complexité du dispositif. Je demande et on est un certain nombre à demander aujourd'hui que les demandes de remboursement soit reporté, repoussé pour qu'on examine la situation des communes concernées sur deux 3 4 ans parce que sinon une aide va déstabiliser encore plus la situation financière de ces communes, c'est pas le but, j'imagine. Merci, cher collègue, la parole est à présent Monsieur babary pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame le Ministre. Mes chers collègues je ne reviendrai pas sur les nombreuses difficultés rencontrées sur le guichet unique aux entreprises par les déclarants en matière de création modification radiations. Tout à l'heure notre collègue Vina. A pu échanger avec vous Madame la Ministre sur ce sujet. Certaines des difficultés rencontrées ont été résolues avec la réouverture partielle d'info. Le dépôt des comptes annuels des entreprises ne bénéficient malheureusement pas de cette réouverture et doit donc être réalisé via le guichet unique. Or, dans le cadre des travaux de la délégation sénatoriale aux entreprises nous avons été alertés par l'Ordre des experts-comptables ainsi que par de nombreux entrepreneurs, au sujet de nombreux bogues et anomalies rencontrées au moment de ce dépôt dématérialisé. Des pièces non-obligatoires, tels que le rapport de gestion des micro-entreprises ou encore la déclaration de publicité peuvent être exigé qui bloque l'examen de ce dossier. Les entrepreneurs rencontrent également des difficultés en raison du format numérique PDF compléter en ligne exigé par la plateforme aussi il existe aujourd'hui une véritable inquiétude concernant l'accomplissement de cette formalité dont le flux devrait augmenter de manière exponentielle. Au cours des mois de mai et de juin. L'absence de réalisation de cette formalité susceptibles d'emporter de graves conséquences pour les entreprises concernées amende ou refus de financement de la part des banquiers. Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer la fiabilité du système. Réfléchissez-vous à la mise en place d'un format de données informatisées tels que cela est évoquée par l'Ordre des experts-comptables d'une manière plus générale, que va-t-il se passer au 1er juillet. Quand le guichet unique reprendra toutes ses missions. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci beaucoup monsieur le sénateur, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Babary, vous avez raison hein c'est une remontée qu'on a sur nos territoires de manière assez simple et sans expertise ministériel La réglementation qui prévoit effectivement que les entreprises soient soumises à cette obligation de dépôt des comptes réalise cette formalité par voie papier soit par voie dématérialisée depuis le 1er janvier 2023. Ce dépôt en ligne se fait exclusivement sur le guichet unique en application de la fameuse loi pacte dont dont on a parlé il il y a quelques instants. Alors quelques chiffres peut être 100.000 dépôts papier environ ainsi que 25.000 dépôts en ligne et franchement les difficultés qui ont pu être rencontrés ont été identifiés. On y retrouve un certain nombre de témoignages que vous venez de rappeler des actions de remédiation ont été initiés cependant une 2ème version de cette procédure simplifiée par rapport à la voix initial a ainsi été ouverte juste là en avril sur le guichet unique de l'INPI. Alors ça a été élaboré avec les experts comptable et les mandataires qui sont les principaux déposants et il faut s'appuyer sur ce qui accompagnent au quotidien. Monsieur le sénateur, je crois que on peut se rejoindre sur ce point elle réduit dû notamment le nombre d'États préalables qui étaient peut-être un peu trop gourmand pour rester. Est rester diplomatique. Sur les propos des étapes qui a mené à des risques d'erreurs directement liés à l'utilisation du guichet parallèlement en lien avec les greffiers également des tribunaux de commerce qui valide ses dossiers de bonnes pratiques ont été élaborés et partagée par les déposants professionnel qui leur permettent de mieux identifier les motifs de rejet. Qui parfois qu'on créé des incompréhensions assez importante et donc améliorer la qualité des dépôts ces actions. Monsieur le sénateur, ont vocation à améliorer l'expérience utilisateur d'une certaine manière de ses déposants pour que le dépôt des comptes en ligne sur les guichets soient franchement une une brève échéance que ça ne crée pas de stress supplémentaire, compte tenu de la situation déjà. À surmonter et on observe d'ailleurs dès l'avoir récemment ouverte et d'ores et déjà un peu plus utilisé par les déclarants. Vous pouvez compter sur la pleine mobilisation du gouvernement pour la mise en place de ce, de, de cette. Nouvelle opérationnalité du guichet unique tout comme vous pouvez compter sur notre vigilance et Monsieur le Sénateur, vu que c'est un sujet qui vous tient à coeur. Je m'engage à ce que le ministre en charge vous fasse un retour sur les étapes à venir. Je vous remercie. Monsieur babary vous pouvez compléter votre question. Madame la Ministre je vous remercie. Cependant, cette affaire de plateformes. Elle dure depuis un moment, j'ai interrogé Bruno Lemaire le 18 juin. Voilà sa réponse. Nous avons laissé l'INPI jusqu'au début du mois de mars, pas plus tard pour que le site soit effectif. Opérationnel. D'accès Direct. J'ai visité avec la délégation aux entreprises que je préside l'INPI le 8 février. Nous avons vu les responsables. J'ai interpellé Olivia Grégoire. Le 22 mars. Lors. Sa réponse ce projet comme tout projet informatique d'ampleur et complexe. Ce que vous dites mais nous serons au rendez-vous fin juin. Je pense que il faut vraiment prendre définitivement la mesure de la difficulté pour les entrepreneurs et l'affaire du dépôt des comptes annuels est très grave puisqu'il y a des blocages des maintenant déjà il faut prendre la tâche des experts-comptables, merci. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame, Colette Mélot pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre agir pour la réduction des inégalités sociales de santé. Est aujourd'hui une priorité des politiques publiques. Mais nous le savons, les personnes en situation de handicap sont potentiellement plus vulnérables et moins réceptives aux actions de prévention. Les campagnes de prévention sont difficilement accessibles aux malentendants dans la mesure où la maîtrise de la lecture ayant été freinée par le handicap peut les mettre en difficulté dans la compréhension des messages de plus les sous ont un mode de communication très visuel qui rend les supports de prévention classique peu adaptée à ce public. Ainsi pour les jeunes malentendants scolarisés public vulnérable aux difficultés multiples. L'accès aux informations santé qu'il s'agisse d'addiction d'alimentation de santé sexuelle de santé mentale d'écrans et de réseaux sociaux de harcèlement scolaire même est un problème massif, et ce quel que soit l'âge. L'information qu'ils reçoivent souvent parcellaires. Parce que peu adaptés à leur handicap. Cela s'explique aussi par le fait que les interprètes sont encore trop peu nombreux. Et que le 114 ou encore Fil Santé Jeunes qui a mis en place un service d'interprètes sont si l'on en croit les jeunes concernés encore trop méconnu. on l'on y ajoute que la lecture et la compréhension sont parfois compliqué l'addiction de ces facteurs a pour résultat un isolement dont les personnes concernées m'ont fait part avec des conséquences psychologiques parfois désastreuses. Le service de santé de l'éducation nationale doit pouvoir interagir avec les jeunes et leurs familles. Les interprètes les codeurs les AESH les services de soins afin de préparer et accompagner les actions de sensibilisation et favoriser l'accès à des supports adaptés Madame la Ministre alors que les déserts médicaux sont une réalité dans notre pays et que la prévention est l'un des défis majeurs de notre politique sanitaire. Comment créer les conditions nécessaires pour que les campagnes diffusées dans les établissements scolaires, puissent être accessible à ce public. Merci. Si cher collègue Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Mélo. On connaît votre engagement pour une école inclusive et pour l'ensemble de ses enfants, qu'ils soient en territoires urbains ou ruraux qu'il soit porteur d'un handicap ou pas et Madame la sénatrice. Vous avez raison, la promotion de la santé à l'école est un essentiel, on ne peut pas dire que l'école c'est l'éducation, c'est la mère des batailles et ne pas accompagner chacun de ses élèves chacun de ses enfants de la même manière on sait très bien que l'école. Qui promeut qui fait la promotion de la santé permet un climat scolaire de qualité et donc d'une certaine manière de rendre tangible quasiment en la promesse républicaine qui est celle de l'égalité mais la réalité elle est là, il y a encore en réalité de grande. De grande difficultés malgré l'objectif de renforcer le pouvoir d'agir des élèves malgré la lutte contre les discriminations liées handicap à l'intérieur de l'école, les élèves sourds comme les autres élèves ont un droit fondamental à l'éducation et ce droit impose au système éducatif, de s'adapter et j'insiste sur le mot ce droit impose que le système s'adapte s'date pour leur offrir les meilleures chances de réussite et une diversité dans leur parcours et pas une limitation. Il y a pas de raison et pour cela la scolarisation d'abord. C'est vrai en classe ordinaire mais aussi en unité. Localisée pour l'inclusion scolaire en unités d'enseignement. La mise en place de parcours de formation pour les jeunes sourds dans des pôles d'enseignement. Pour jeunes sourds sont en développement croissant cependant concernant l'accès aux informations écrites et notamment à la lecture, c'est ce que vous avez souligné un programme d'enseignement bilingue en langue des signes. Et la langue française écrite devrait être prochainement. J'ai fondé énormément d'espoir. Et je, je sais que vous y voilà vous vous suivez ça de très près. Madame la sénatrice, l'apprentissage. De la lecture pour tous les élèves sourds est un enjeu fondamental pour l'expression d'une citoyenneté éclairée également et l'enseignement. De la LCF. Et en LCF par les professeurs garantit. L'éducation à la santé aussi. Hein aux élèves en situation de surdité enfin à la transposition de la direction européenne. En droit français sur l'accessibilité native des livres numériques va je crois dans le sens évidemment de cette accessibilité universelle pour l'ensemble des élèves, madame la sénatrice je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pour que ça soit fait dans rapidement. Merci, madame la Ministre, la parole est à présent madame Nadège avait pour sa question. 430.000 enfants, 100.000 de plus par rapport à 2017 qui bénéficie d'un parcours adapté dans les écoles avec des ALSH à leurs côtés. Je veux saluer ce matin l'engagement de ces professionnels, de même que le soutien des pouvoirs publics à cette nécessaire politique d'inclusion. Cependant, les 120.000 personnes mobilisées correspondent dans les faits à 80.000 équivalents temps plein. Beaucoup n'ont pas de contrat plein et ont par conséquent des rémunérations plus faibles. Cela doit nous interpeller avec cette question comment parvenir à proposer des 35 heures hebdomadaires. Cette problématique a donné lieu à une prise de parole du président de la République il y a un mois. Il a justement rappelé que les vraies difficultés c'est d'avoir un temps complet. Ma question portera sur ce point et elle fait suite à une première réunion avec le cabinet du ministre en septembre dernier interpellés début 2022 par de nombreux élus finistériens sur les difficultés à recruter recruter et à maintenir en poste ces professionnels notamment du fait de l'articulation difficile entre les temps scolaires et périscolaires. Il semble que l'une des réponses pourraient être en effet la mise en oeuvre d'un dispositif global afin d'éviter d'une part la rupture dans l'accompagnement des enfants et d'autre part garantir la continuité et la cohérence des modalités d'intervention des AESH avec l'objectif de consolider leur contrat pour faire suite à la décision de 2020 du Conseil d'État la proposition spécifique de mise en oeuvre d'un conventionnement de mise à disposition des AESH recrutés par l'Éducation nationale lorsque leur présence est requise par sur les temps périscolaires pourrait s'avérer être une réponse pertinente alors qu'il faut déterminer la meilleure formule juridique, de même que la solution administrative la moins lourde possible pour les collectivités territoriales et pour l'État. Je souhaite savoir où en sont les avancer sur cette question, je vous en remercie. Madame la ministre, votre réponse est attendue. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice avait. De la même manière, je connais votre engagement pour les enfants en situation de handicap et en réalité pour une école inclusive plus largement madame vie je vais sortir de de mes notes, pour une raison toute simple. Aujourd'hui, l'accompagnement des AESH est absolument nécessaire pour garantir l'égalité et l'inclusion des élèves en situation de handicap. La réalité c'est qu'effectivement le Conseil d'État a rappelé dans sa décision de novembre 2020 qu'il revient pas à l'État d'organiser financièrement mais aux collectivités. Cependant, cependant, c'est quoi la priorité des priorités c'est l'intérêt de l'enfant, c'est l'accompagnement des familles. Donc évidemment nous avons des points de droit, je vous l'accorde mais plus que jamais comme pour les accueils collectifs de mineurs pour, comme pour le périscolaire, comme pour l'extra-scolaires, nous avons des métiers qui sont des métiers de vocation et sur lesquels il faut d'une certaine manière concret hé bien une sécurisation. Un peu moins de précarité pour créer de l'attractivité à ESH animateurs éducateurs et qu'est-ce qu'on voit arriver, hé bien on voit des métiers pour qui. Et, me dit-on, dans lequel on reste pas où on reste peu alors même qu'ils sont essentiels, si on croit à la complémentarité entre l'éducation formelle et l'éducation informelle, c'est-à-dire l'apprentissage l'instruction des fondamentaux pendant les heures de classe et en même temps, pendant le temps Méridien ou en dehors du temps Méridien finalement le développement des fameuses compétences transversales nécessaires. À une bonne scolarité, alors nous avons besoin d'avoir un trait d'union, je sais que le cabinet du ministre de l'Éducation nationale à la suite des annonces du président de la République s'est particulièrement mobilisée pour annoncer que dans les centres de loisirs, les enfants de 3 à 17 ans verront un bonus périscolaire soutenue par les CAF. Nous sommes en pleine négociation des causes de la CNAF, ce n'est pas anodin et j'insiste sur ce point peut-être plus spécifiquement. Parce que ce sera un rendez-vous qui va conditionner les 5 prochaines années sur cet accompagnement-là et donc l'accompagnement des jeunes, des enfants, des jeunes et en réalité également des adolescents sur tous les temps d'apprentissage madame les sénatrices à ESH. Animateur accompagnateurs sont aujourd'hui des. Des pépites en réalité de notre système. Hé bien d'éducation informelle, nous avons besoin de leur proposer des formations complémentaires des métiers à temps complet plus attractif et qui paye mieux parce que si on nomme les choses on trouve des solutions. Je vous remercie. Merci madame la ministre. La parole est à présent monsieur Olivier Rickman pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de la fonction publique Stanislas Guerini. Mais vous ne pouvez ignorer ce sujet sur lequel j'ai sans succès manifeste interrogé le gouvernement à plusieurs reprises et qui fait l'objet depuis quelques semaines une couverture médiatique remarquée le 6 mars dernier j'adressais d'ailleurs un courrier à votre collègue, le ministre Olivier Dussopt, qui la veille dans l'hémicycle, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les retraites s'était engagé à trouver une solution avant l'été pour ces professeurs, victime d'un véritable cafouillage administratif. Ce courrier a finalement été transmis au ministre-Guérini par le cabinet du soap et par moi-même. 30.000 enseignants seraient concernés. Ils ont en commun d'avoir suivi au début des années 90. Une formation à l'IUFM au cours de celle-ci, la loi leur permettait de bénéficier d'une allocation censée être pris en considération dans le calcul pour leurs droits à la retraite. Or, le décret d'application de cette loi du 26 du 26 juillet 1991, n'a jamais été publié, cette disposition n'est donc actuellement pas appliqué, c'est-à-dire que les trimestres acquis par l'enseignant au cours de la période de formation ne sont pas comptabilisés. Dans une réponse datée du 30 mars 2023. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Conscient de la gravité de la situation, écrit que celle-ci ne peut pas perdurer et que des travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions apportées elle les mettre en oeuvre dans les meilleurs délais. Madame la Ministre, vous l'aurez compris ma question est donc simple à quelle date votre gouvernement entend-il publié le texte réglementaire manquant. Serez-vous en mesure de respecter l'engagement pris par votre collègue Olivier Dussopt, de faire entrer en vigueur la disposition avant l'été. Je vous remercie. Madame la ministre, votre réponse. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Hitman. Votre question a le mérite d'être particulièrement. Ce qui amène à une réponse plutôt clair.

à. Répondre à cet engagement qui est pris pour plusieurs raisons. Un engagement qui est pris au banc hé bien engage ça fait partie un peu de ses essentiel de confiance dans notre dans notre dans notre en charge. Des travaux avec le ministre-Stanislas Guérini, Guérini. La mise en place de l'article 14 de la loi du 26 juillet 91 et nécessaire est engagé.

dès qu'il sera transmis ce qui est certain monsieur le sénateur, pour pas rajouter cafouillage a cafouillages cafouillages. Hérité c'est que. L'article 14 de du 26 juillet 91. Il n'y a pas de raison qu'il continue à s'appliquer. Il y a inégalité, donc il faut une réponse à une réponse le plus rapidement possible. Je vous remercie. J'collègue, vous avez un temps de parole supplémentaires. Merci monsieur le président. Merci, madame la Ministre, de votre réponse qui ne la satisfait pas effectivement. L'engagement a été pris à 30 ans réitérée par le Ministre Dussopt il y a il y a 3 mois réitérée par le ministre et l'éducation nationale et par vous-même ce matin. Avant l'été s'est engagé le Ministre Dussopt. 30.000 enseignants vous ont entendu ce matin moi également. On suivra la réponse et on y reviendra s'il le faut. Merci.

Monsieur le président, madame la ministre. Alors c'est vrai que, ma question s'adresse aussi à madame la ministre de la culture puisqu'elle concerne les difficultés en cours et à venir pour les spectacles subventionnés et en particulier les festivals. Donc, en raison d'une d'une succession de problèmes liés au contexte mais pas que les spectacles doivent réduire leur taille pour éviter une une déroute financière ainsi la la récente poussée inflationniste avec en particulier l'augmentation des prix de l'énergie, qui ont été multipliés par voire par quatre a conduit à des situations compliquées les saisons été raccourci et on déplore beaucoup d'annulations. Le Syndicat national des scènes publiques a annoncé plus de 100.000 spectateurs perdus pour cette année. Où en est-on réellement. Il nécessaire d'assurer un meilleur avenir dans le domaine du spectacle vivant alors qu'il faut aussi compter avec l'augmentation du point d'indice et des salaires des intervenants, les conventions collectives qui qui renchérissent les coûts et les charges pour les festivals. D'autres facteurs plus anciens contribue à l'asphyxie budgétaire comme l'empilement des missions et les exigences classique d'écoulement découlant des cahiers des charges, donc la médiation culturelle, l'éducation artistique, les projets avec les établissements scolaires ou pénitentiaire quant au soutien des collectivités territoriales. Il ne suffit plus à couvrir les charges fixes. Pourtant, le 9 février dernier des aides exceptionnelles ont été annoncées pour soutenir les structures les plus en difficulté confrontée notamment à la à la hausse des prix de l'énergie donc j'aimerais également savoir où l'on en est ainsi dans le Grand-Est, ont donc ma région. On parle de 17 équipement et structures qui vont recevoir une aide différenciée, qui va de quelques millions d'euros à 70.000 euros mais il n'y a pas davantage de précisions. Donc si l'on veut assurer la pérennité du festival. Il faut éviter évidemment de toucher aux tarifs donc la question de la survie interroge et pose en réalité la question de la place que vous que l'on veut donner à la culture dans notre pays. Merci, cher collègue, la parole est à la ministre. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Joseph je connais de loin votre attachement au spectacle vivant et à la vie culturelle sur votre territoire. Mais plus largement c'est vrai dans notre pays. Ça fait partie de ce génie français ça fait. La la culture sa vivacité et même son caractère particulièrement populaire permet de faire, hé bien j'aurais dit d'une certaine manière, je veux dire le peuple que nous sommes et son accompagnement est nécessaire, vous évoquez l'enjeu des festivals. Il se trouve que c'est un sujet qui touche aussi particulièrement l'ouest et donc mon territoire plus de 7000. En particulier l'été et votre département en compte un certain nombre en préparant la question. La ministre de la culture m'a rappelé naturellement le Cabaret Vert. Au Festival mondial des théâtres de marionnettes et c'est vrai que. En relisant et en préparant la réponse. Ça donne plutôt envie de venir. Le soutien financier de la part du ministère de la culture est important effectivement 800 festival soutenu en 2022, 31 millions d'euros qui viennent en complément de l'action du Centre national de la musique apporte son aide. en relevant. De la taxe des spectacles. Il a ainsi soutenu 155. Festival de musique en 2022 pour 4 millions d'euros. Cependant l'inflation. Ça, c'est notre quotidien et c'est la réalité qui touche tout le monde. Le coût de l'énergie aussi. Et le gouvernement a été au rendez-vous au-delà des aides transversales mises en place par le ministère de l'économie. Ma collègue Rima Abdul-Malak a annoncé le 1er mars dernier effectivement des aides exceptionnelles. Vous les avez souligné madame la sénatrice, ça touche 17 structures en particulier sur votre territoire la de la Comédie de Reims, en passant par leur caisse nationale de Metz ou encore la Scène nationale de Mulhouse Mulhouse chaque structure aider s'est vu communiquer par la Drac le montant à louer des précisions si vous le souhaitez-vous pourront être transmises puisque c'est le sens de votre de vente et au delà à madame la sénatrice le le ministère de la culture travaille de façon étroite et en concertation avec l'ensemble du secteur du spectacle vivant pour relever ces défis économiques et environnementaux qu'ils rencontrent parce que nous en avons besoin pour aussi retrouver cette espérance et cet élan dont nous avons en réalité la conditionnalité. Je vous remercie madame. C'est Mario. Vous avez quelques secondes. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques secondes parce que c'est vrai qu'on partage cette préoccupation où il faut vraiment changer le modèle économique des festivals et il y a une question aussi que je n'ai pas posé. C'est la question de comment faire revenir les jeunes parce qu'on a quand même un souci là-dessus et, bien entendu. Vous êtes les bienvenus à nos 2 grands événements majeurs de cet été puisqu'on a le Festival international des théâtres de marionnettes en septembre et le festival du Cabaret Vert et comme ça on pourra discuter concrètement avec les acteurs du territoire. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Laurent Somon pour sa question. Monsieur le président, madame la Ministre, chers collègues. Les grands événements sportifs internationaux en France. Ce sont des événements utile au pays, pour son rayonnement et son économie, mais aussi des sujets d'engagement de nos territoires par les ressources de l'accueil qu'elle propose et par l'engouement qu'elle suscite, voir les vocations il les désirs de pratiques qu'elle révèle. Permettez-moi quelques poignées de semaine des chiffres d'olympiques de 2024, de rappeler notre projet de sport pour tous dans tous les territoires de l'Hexagone avec les compétitions organisées dans une dizaine de villes. Le reste du territoire et plus éloigné de ces grands moments de fête pour les populations et donc l'accompagnement au développement et à soutenir comme par exemple la réhabilitation des gymnases affecté au collège en particulier. Et puis éviter surtout la désillusion d'un événement sportif qui pourrait permettent justement de générer des équipements. L'Agence nationale du sport intervient dans l'élaboration et le déploiement de programmes d'intervention, avec l'objectif des politiques sportives en cette période. Je demande au gouvernement quels moyens et quelles Z quelles actions seront portées par la NS et la direction des sports en faveur des équipements sportifs en milieu rural et en particulier pour les gymnases dans les zones les plus retranché qui en dehors des sites d'accueil des Jeux olympiques et ceux des équipements au rayonnement large des grandes villes ne sont pas souvent retenue dans les programmations et si elles reposeront sur un juste équilibre de l'offre des disciplines et des infrastructures le permettant. Dans tous les territoires des départements de métropole et d'outre-mer. Merci cher collègue. Madame la ministre, nous vous adressons nous donnons la parole, Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs Madame. Monsieur le Sénateur saumon vous interroger effectivement la ministre des Sports et elle ne pouvait pas. Présente mais m'a transmis sa réponse puisque. Vous avez raison sur un point absolument essentiel. Les Jeux olympiques qui arrive dans une poignée de semaines pour reprendre votre expression. En réalité c'est un grand rendez-vous mais c'est un rendez-vous qui doit permettre d'inclure tout le monde et de laisser un héritage et pour le coup pour que ce soit un grand événement populaire, alors il doit irriguer. Il doit irriguer le sport pour tous, il doit irriguer les familles les plus jeunes et permettre à chacun est bien de le vivre au plus proche. L'état les mouvements sportifs, les collectivités territoriales, tout le monde franchement monsieur le sénateur s'est retroussé les manches pour faire que ce grand rendez-vous soit une réussite. Le les les engagements de la NS sont fondés sur 2 piliers la haute performance et le développement de la pratique sportive pour tous. À ce titre, la mission de corriger les inégalités.

Pour un montant de subvention de plus de 117 millions d'euros plus particulièrement 58% des rénovations d'équipements au titre du plan de relance 2021 2022 ont bénéficié également aux territoires ruraux pour un montant de 34 millions d'euros en parallèle la mise. En place la première année du déploiement de 5000 terrains de sport, lancée par le président de la République en octobre 2021. À bénéficier prioritairement également aux zones rurales qui ont fait l'objet de plus de 70% des équipements financés pour un montant de 51 millions d'euros. aujourd'hui on parle de millions, on parle de plusieurs milliers d'équipements sportifs. Je crois que ce qui compte c'est quand. Hé bien on trouve les voies et moyens pour accompagner le développement de en réalité de terrain de sport de parler vous parliez de gymnase quand les élus locaux quand l'état et la NS se retrouvent autour de la table et quand parfois la ferveur d'un territoire a su trouver réponse je vous remercie.

Merci, monsieur le Président Madame la Ministre j'appelle votre attention sur le complément de traitement indiciaire au sein des établissements et services médico-sociaux autonomes. a été institué pour les personnels des établissements de santé pour répondre aux enjeux de reconnaissance et de valorisation du secteur. Pourtant, le personnel des filières administratives, logistiques et techniques dans les établissements publics déco sociaux autonomes qui ne sont pas rattachés à un service hospitalier sont exclus de ce dispositif. Ainsi, les agents des services hospitaliers, les personnes qui travaillent auprès des résidents et des personnes handicapées dans la maison d'accueil spécialisée le foyer Claire situé à en de l'eau dans mon département sont exclus de ce dispositif. Il relève pourtant de la fonction publique hospitalière. À contrario, le personnel des filières administratives, logistiques et techniques qui effectuent les mêmes tâches dans des Ehpads non rattachés bénéficient de ce complètement de traitement indiciaire. la directrice qui gère 2 établissements perçoit ainsi moitié de cette prime pour ses missions au sein du Nepad. Avec à contrario rien pour les mêmes missions dans la masse dans de l'eau, il y a une véritable injustice et l'iniquité de manière générale. Il reste en France encore 3000 agents de la fonction publique hospitalière privée de ce ces pays ainsi je souhaite avoir tous les éclaircissements nécessaires pour expliquer cette différence de traitement entre une maison d'accueil spécialisée public non rattachés pour lesquels le personnel des filières administratives, logistiques Nobel. Je ne suis pas de ce 7 alors que les agents du même grade qui exerce les mêmes fonctions dans un Ehpad non rattachés bénéficient de cette revalorisation et je souhaite donc savoir si cette situation sera régularisée. Et selon quel motif les professionnels concernés n'ont pas été revalorisés au même titre que les autres agents de la fonction publique hospitalière. Merci, cher collègue, la parole est à madame la ministre Firmin Le Bodo. votre fournir les éléments suivants, en réponse à votre interrogation. L'attractivité des métiers du secteur sanitaire, sociale et médico-sociale est au 1er rang de la feuille de route du gouvernement nous entendons agir sur l'ensemble des d'attractivité avec une action déjà déterminé sur la revalorisation de ses métiers mais je pense aussi aux enjeux d'accès à la formation continue d'amélioration des conditions de travail ou encore de lutte contre la sinistralité vous avez justement rappelé les mesures fortes prises par l'État aux côtés des départements en faveur des rémunérations à la fois au titre du Ségur mais aussi de la motion dite Lafourcade avec près de 700.000 salariés concernés. L'ensemble de ces mesures a fait l'objet de travaux préparatoires qui ont largement associés à chaque fois les acteurs concernés, avec des gains d'attractivité réelle pour certains merdier en tension. Pour autant, il convient de poursuivre les actions menées à destination de l'ensemble des professionnels. Pour cela, il convient d'arriver aux côtés des représentants des employeurs et des salariés à la construction d'une convention collective unique pour le secteur social et médico-social. C'est la condition d'une revalorisation durable des parcours professionnels de l'ensemble des personnels du secteur y compris techniques et administratifs l'état et l'association des départements de France ont annoncé le 18 février 2022 qu'ils sont prêts à mobiliser 500 millions d'euros pour faire aboutir ces travaux. Les discussions sur l'augmentation des rémunérations et notamment les plus bas salaires doivent prendre leur place dans le cadre de cette convention collective unique. J'ajoute que l'enjeu de l'attractivité de ces métiers ne se résume pas à ses seule revalorisation c'est l'ensemble de la politique que nous menons, qui doit nous permettre de reconnaître la pleine valeur des professionnels mobilisés chaque jour aux côtés de nos concitoyens les plus vulnérables. Si Madame la Ministre, chers collègues. Vous pouvez compléter votre question. Oui ben je je note Madame la Ministre je vous remercie pour la réponse que vous nous avez lu. Qui vient de du ministre concerné mais je note ce que je n'ai pas de réponse à ma question, est ce personnel attendent cette revalorisation merci. La parole est à présent Madame Valérie Boyer pour sa question. Monsieur le Président Madame la Ministre. Je voudrais vous alerter vous alerter, parce que depuis plusieurs mois, la CNAM a annoncé son désir de reprendre en matière de dépistage des cancers. pilotage des invitations de la population sous prétexte qu'elle permettrait de meilleurs résultats de participation et qu'elle ferait des économies. Pourtant il n'en est rien puisque les cendres de coordination s'inquiète d'une forme de nationalisation du dépistage sans garantie d'une amélioration du taux de participation depuis 2019. Ils assurent pourtant cette mission d'envoi d'invitation en lien avec les ARS et les directions de la coordination et de la gestion du risque. Il joue un rôle pivot est essentiel de coordination. Malheureusement, l'assurance maladie en prenant cette nouvelle mission d'invitation malgré l'avis de tous les professionnels et élus locaux indique également qu'elle ne communiquera pas assez Centre de dépistage les fichiers des populations c'est beaucoup de brutalité madame cela impliquera que le suivi ne pourra pas être assurée par ses cendres de dépistage, cela sera lourde de conséquences en induisant une perte de qualité du suivi médical et donc une dégradation du système de santé au profit d'une seule campagne l'invitation. Pourtant, ces cendres qui bénéficient d'une visibilité locales sont prêts à orienter la majeure partie de leur activité autour de la prévention mais aussi souhaite d'une part s'investir pour lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé mais aussi optimisé la prise en charge des personnels à des personnes à risque élevé de cancer, alors pourquoi une telle précipitation de la part de la CNAM alors que rien ne peut garantir que cette opération va faire monter la participation pourquoi désorganiser ce qui fonctionne très bien depuis d'ailleurs les années 90 aussi. Envisagez-vous de revenir sur ce choix qui impactera demain lourdement la qualité des dépistages des cancers en France qui fera perdent qui fera perdre des chances au malade et qui placera la France, en dehors des indicateurs de qualité des dépistages organisés en Europe. Si cher collègue, la parole est à madame la ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. Le ministre François Braun regrette de ne pouvoir être présent il m'a prié de vous fournir les éléments suivants, une politique efficace de prévention primaire et de dépistage est essentielle pour lutter contre le cancer, c'est une priorité de notre action 3 programmes de dépistage organisé ont été mises en place pour le cancer du sein colorectal et du col de l'utérus. La stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021 2030 portent également des actions ambitieuses notamment pour améliorer l'accès au dépistage. Une nouvelle feuille de route des dépistage organisé des cancers priorité dépistage a été annoncée en décembre 2022 par la Première ministre avec une organisation rénovée. Des dépistages et des premières mesures d'évolution des missions des centres de coordination des dépistages des cancers. Les serres le transfert début 2024 à l'assurance maladie du pilotage des inventeurs d'action à participer à un dépistage organisé le recentrage des missions confiées Auxerre CDC sur leur mission essentielle de suivi des résultats des programmes de dépistage organisé d'information et de formation des professionnels la mobilisation systématique de réparation d'aller vers par la caisse d'assurance maladie mobilisant tous les acteurs de prévention dont les serres CDC sous pilotage des ARS cette nouvelle organisation doit contribuer à augmenter la réalisation des dépistages organisés pour mener à bien ses travaux la DGS a annoncé le 19 janvier dernier le lancement en lien avec l'assurance maladie de plusieurs chantiers préparatoire sur les invitations et là les Verts en 2023, des représentants des CDC sont évidemment associée des premiers jalons de la future organisation ont déjà pu être mises en place sur le Champ de l'aller vers la poursuite des missions des CDC a ainsi pu être confirmée en lien à être les autres acteurs de prévention et sous coordination des ARS, les points d'attention que vous soulignez sont bien identifié par nos services dans la mise en place de cette nouvelle organisation nous restons par ailleurs vigilant à l'équilibre financier et aux moyens qui seront alloués Auxerre CDC pour mener à bien leur mission. J'invite donc les serres CDC à pousuivre leur contribution aux travaux en cours afin de réunir ensemble à la mise en oeuvre de cette. Nouvelle feuille de route. vous voyez. Il vous reste un temps pour répondre. Non. Un mini. J'ai toujours pas compris pourquoi vous casser ce qui fonctionne aujourd'hui ça fonctionne bien, c'est depuis les années 90 et c'est effectivement, ça concerne les 3 cancers le cancer du sein, le cancer que Laurel. Et le cancer du col de l'utérus. Vous savez bien que les campagnes de SMS auprès des publics précaires, ça ne fonctionne pas et aujourd'hui. La question est la suivante, pourquoi se précipiter pour casser ce qui fonctionne, contre l'avis de tous les professionnels de santé et élus locaux, il y a beaucoup d'inquiétude. Je ne voudrais pas qu'il y ait beaucoup de pertes de chance avec cette nouvelle façon de travailler parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. La parole est à présent président de l'âtre qui remplace notre collègue Cabanel qui a la parole. Oui, merci Monsieur le Président Madame la Ministre, mes chers collègues je pose effectivement cette question en en lieu et place de mon collègue sénateur Henri Cabanel, pour qui j'ai une pensée de prompt rétablissement qui s'est, il s'est blessé sur son exploitation viticole Henri Cabanel souhaité attirer votre attention, madame la Ministre, sur les inquiétudes des infirmiers libéraux quant à leur situation qui se dégrade pendant la Covid. Ils ont prouvé qu'ils incarnaient des acteurs indispensables tout du long du processus observé pendant la crise sanitaire dépistage soins vaccination. De plus, ils ont démontré leur faculté d'auto-organisation pour coordonner un centre de 6 nations et intervenir pour tester soigner et surtout. En tous lieux à domicile dans des bateaux dans des bus ou des tentes dans les écoles ou encore dans des centres de sans abris, tout en continuant à prendre en charge leurs patients habituels tout au long de l'année, ils se retrouvent contraints de travailler les week-ends. En plus de la semaine pendant leurs congés, voire même pendant leur temps de pause. Alors face à cet engagement sans faille, une revalorisation de leurs actes et de leurs indemnités kilométriques est-elle car les actes médicaux infirmiers les fameuses amis sont bloquées depuis l'augmentation de 15 centimes obtenus en avril 2009 et leurs indemnités kilométriques sont inférieures à celles d'autres professionnels de santé, ce qui est injuste car la hausse de carburant étant identique pour tous. Je vous remercie. La parole est à vous, madame la Ministre. été moi-même vendredi avec une infirmière libérale pour faire sa tournée du matin s'agissant de la rémunération des infirmiers libéraux, la mise en place du bilan de soins infirmiers bé ici en 2020 à rénover le modèle de facturation des actes forfaitaire journalière adaptée à l'état du patient âgé complexe le BSI a connu un succès important auprès de la profession. Ainsi l'avenant numéro 8 de janvier 2022 à la convention des infirmiers libéraux, prévoit un doublement de l'investissement sur le ici sur 2022 1024 avec un montant de 217 millions d'euros contre 122 millions d'euros prévus initialement. Le dispositif du BSI vise également à améliorer la prise en charge et l'accès aux soins des patients notamment par le développement et la coordination pluri-professionnelles et l'investissement dans la dans la prévention. Si le mener pour le du BSI a été décalée en raison d'un impact financier supérieur aux prévisions cette réforme du mode de financement des actes infirmiers demeure pertinente aussi là l'avenant numéro 9 de juillet 2022 comporte 22 millions d'euros de rémunération notamment pour les infirmiers en pratique avancée sur les indemnités kilométriques une révision du mode de calcul des indemnités kilométriques est déjà intervenu en 2019 et l'assurance maladie à revaloriser pour la seule année 2022, les indemnités kilométriques des infirmiers libéraux pour compenser la hausse du coût du carburant. Cette mesure c'était cumulées avec les remises de l'État accessible à tout conducteur. Plus largement, en tant qu'acteur majeur de l'organisation des soins, sur le territoire en raison de leur effectif et de leur polyvalence les infirmiers libéraux et les conditions de travail occupe une place centrale dans les travaux de transformation du système de santé que nous menons, nous avons lancé une mission conjointe de l'IGAS et de lisier ESR sur l'évolution de la profession et de la formation infirmière qui préconise des transformations sur ces 2 champs pour mieux valoriser et accompagner les infirmiers des leurs études nous travaillons notamment l'intégration du mentorat dans les formations à l'encouragement et la meilleure reconnaissance du tutorat et au déploiement des dispositifs quelque les cordées de la réussite. Merci madame la ministre et la parole est à nouveau à la présidente de l'autre. Oui, merci Monsieur le Président, je vous remercie. Madame la Ministre pour votre réponse détaillée par ce qu'il y a effectivement urgence en raison des difficultés que je viens d'évoquer. Près de 60 infirmier sur 100 envisage de quitter leur profession d'ici à 5 ans face à une population française vieillissante. Il faut absolument arrêter cette hémorragie et accéder aux revendications de la profession que j'aurais pu également Je pense à la revalorisation des lettres-clés de leur nomenclature ainsi qu'à une meilleure prise en compte de la pénibilité de la profession pour les droits à la retraite, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame ah nous allons, pour ce qui est. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre le centre hospitalier d'Ardèche méridionale souffre d'une pénurie médicale d'autant plus qu'il ne dispose pas des moyens de CHU. Mais sa situation est à ce point critique que le service des urgences et depuis le premier avril fermé le soir et la nuit. Si bien que dans ce territoire à l'écart des autoroutes des gares où déjà les secours mettent de plus en plus de temps à intervenir. Les prises en charge s'effectue dans des hôpitaux éloignés. Ainsi les blessés nécessitant une radio se retrouvent réorienter d'un département à l'autre. À moins que celle-ci ne soit repoussée au lendemain matin. Conséquence, l'état du patient s'aggrave ou faute d'imaginer d'imagerie médicale des soins inadéquats lui sont prodigués depuis longtemps la position géographique d'Aubenas est un frein pour le recrutement des médecins et notamment celui des indispensable intérimaire à présent c'est une tension n'est plus tenable. C'est la question de l'égalité devant la survie en cas de d'accident qui se pose. Faudrait-il une prise en charge trop tardive, conduisant au drame, pour que les pouvoirs publics réagissent aujourd'hui 100.000 personnes sont concernées. Cet été, ce seront 300.000 personnes venues pour la saison estivale et pratiquant des loisirs facteur d'accidents et de blessures qui soignera ses patients et dans quelles conditions. Madame la ministre allez-vous permettre la réouverture des urgences de nuit de l'hôpital d'Aubenas pour cela. Seriez-vous prête à réquisitionner des médecins au niveau régional et du fait de la situation d'exception géographique d'Aubenas. Êtes-vous prête impliquer la réserve sanitaire. Si cher collègue, vous avez la parole. Madame la ministre. Merci Monsieur le Sénateur. Madame la sénatrice vous m'interrogez sur la situation du centre hospitalier d'Ardèche méridionale 10 charme. Des mesures ont été engagés de longue date par l'ARS pour soutenir ce territoire financement de postes d'assistants à temps partagé avec le CH de Valence. Financement de la régulation PDSA en SAMU de journée financement d'infirmières. Pour les transports inter-hospitalier depuis début avril, les difficultés structurelles de recrutement de l'établissement ont conduit à la fermeture des urgences de la nuit en privilégiant le maintien du SMUR sur le territoire, les urgences vitales et il faut le dire sont donc assurés et prise en charge au sein du charme. La nuit même si l'affluence estivale dans le sud de l'Ardèche, n'est pas encore au plus haut niveau cette fermeture partielle peut être de nature à générer des inquiétudes et des tensions. C'est pourquoi l'ARS avec les différents acteurs mettent en place un plan d'action portant sur 3 axes principaux, l'offre de soins urgents, volonté de doubler la ligne de la maison médicale de garde détendre les plages d'ouverture, voire d'ouvrir des maisons médicales de garde éphémère dans les zones les plus touristiques. L'optimisation des transports sanitaires avec la mise en place d'une seconde ligne transports sanitaires urgents pré-hospitalier optimiser la mobilisation de transport sanitaire afin d'économiser les sorties du SDIS. L'évitement des passages aux urgences ou les sorties SMUR communication sur le bon usage du recours aux urgences équipé le SDIS en matériel de biologie embarqué cartographier les ressources des médecins effecteur de la PDA Par ailleurs, depuis le 1er mai est mise en place et financés par l'ARS. Un dispositif de gardes postés du SDIS avec des infirmiers formés au protocole d'urgence qui fonctionne sur la zone de Beaune à la réussite de ce plan se fera par la mobilisation collective des acteurs de santé libéraux et établissements. Sur la réforme de l'intérim pour accompagner ces solutions locales comme le plan travaillée par les acteurs d'Ardèche méridionale. Le ministère de la Santé a mis en place des outils comme la majoration de la prime de solidarité territoriale qui rémunère les praticiens qui prêtent main forte dans les établissements en difficulté dont l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le saisi, je le répète, la permanence des soins sera assurée partout grâce à cette notions organisationnelles travailler localement, notre hôpital et renforcer à long terme par cette réforme et les autres transformations que nous menons. Merci ma la mentale on vous avez la parole. Merci, madame la Ministre j'entends bien votre réponse, mais je vous demande vraiment de mesurer qu'avec cet éloignement des CHU et avec cet enclavement les difficultés de l'hôpital de d'Aubenas sont vraiment accru. On fait face à un personnel soignant épuisés et une population qui souffrent de ce climat anxiogène. Donc, n'attendons pas, je le répète, un drame est vraiment un service continu des services d'urgences de l'hôpital d'Aubenas s'impose. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Philippe mouiller pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame le Ministre. Le projet de réforme relatif aux dispositifs médicaux, et notamment aux aides à la mobilité suscite des inquiétudes auprès des personnes en situation de handicap en ce qu'ils remettent en cause notamment la liberté de choix de l'utilisateur. Concernant les fauteuils roulants. Ainsi l'utilisateur n'aurait plus le choix de la modalité d'acquisition du produit, à savoir acheter du matériel neuf ou remis en bonne état d'usage ou bien loué sur une courte ou longue durée. Ce choix serait laisser non plus à l'utilisateur mais aux prescripteurs. Concernant la réforme de la nomenclature des véhicules pour personnes handicapées du titre IV de la liste des prestations et produits remboursables par l'assurance maladie. D'autres dispositions inquiètent également les usagers. Les modalités de restitution du fauteuil roulant, les délais entre deux renouvellement de prise en charge et la question essentielle du niveau de la prise en charge de chaque fauteuil roulant notamment au lendemain de l'annonce du plan de la République. Par ailleurs, les représentants des personnes en situation de handicap appellent de leurs voeux une rectification de la définition de la remise en bonne état d'usage d'un dispositif médical. Il reste d'ailleurs toujours dans l'attente de la programmation d'une réunion de consultation d'un futur récré relatifs notamment au RB UE cette réunion étant promise depuis plusieurs semaines. Les récentes annonces du plan de la République lors de la dernière CNH et du gouvernement suscite de la satisfaction mais également des interrogations. Les personnes attendent que le remboursement intégral des fauteuils roulants annoncée pour 2024 se. Par un remboursement de tous les modèles de fauteuils sans reste à charge et non pas une extension du 100% santé au fauteuil roulant aussi Madame le Ministre je vous serez recoller, sorte de bien vouloir me préciser les suites que vous entendez réservé aux légitimes demandes exprimées par les personnes en situation de handicap. Je remercie. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur Philippe mouiller. La réforme des dispositifs médicaux, et notamment des aides à la mobilité était nécessaire afin de compléter l'offre de fauteuils rembourse remboursé par la Sécurité sociale. Une évolution était attendu pour répondre à la problématique du reste à charge pour les fauteuils roulants les plus spécifiques pour ces derniers, 60.000 personnes en situation de handicap ont encore plus de 5000 euros de reste à charge actuellement les contraintes financières pour les personnes pour lesquelles le fauteuil roulant et le prolongement du corps conditionnent leur choix de fauteuil roulant. Ce choix ne devrait pourtant pas être un choix par défaut. C'est pourquoi nous avons engagé une évolution et un travail avec toutes les parties prenantes, notamment les associations l'objectif hé bien meilleur équipement pour les personnes en situation de handicap et en particulier pour les besoins les plus spécifiques. Concernant le remboursement d'un fauteuil roulant à l'achat ou en location, il se fait sur prescription. La responsabilité du prescripteur implique un dialogue avec la personne en situation de handicap et le Coz échéance ses proches. Demain les possibilités seront élargis avec la liberté de choix des modalités d'accès. Aujourd'hui, elle concerne uniquement l'achat et dans de rares cas, la location de courte durée. De plus, un essai jusqu'à une semaine du modèle le fauteuil roulant pressenti sera possible concernant le travail sur la nomenclature il suit le processus défini pour les dispositifs médicaux avec plusieurs étapes de consultation et de co-construction. La consultation publique par la Haute Autorité de Santé a permis de préciser la nomenclature. La version définitive du texte est en cours de finalisation avec les apports des associations. Enfin le réemploi des aides techniques permettra de mieux servir l'ensemble des usagers notamment ceux ayant une utilisation temporaire des fauteuils roulants. Dans ce cadre des préoccupations écologiques sont partagés par tous, enfin le décret en consultation auprès de la Commission européenne permettra d'apporter toutes les garanties quant à la sécurité et à la performance des fauteuils roulants remis en bonne état d'usage en complément, une norme mais également travailler avec l'Afnor monsieur sénateur, vous pouvez compter sur notre volonté d'obtenir pour les personnes handicapées, un meilleur équipement. Madame la Ministre Monsieur mouillé. Il vous reste le temps de répliquer. Oui merci Madame la Ministre merci de nous rappeler leur engagement du gouvernement il y a pas de doute. Par contre vous n'avez pas répondu ni à ma question du reste à charge et du montant, est-ce que les 5000 euros seront pris en charge. Non, ni non plus des problématiques du libre choix puisque vous avez posé le débat mais sans réponse directe. à la fois la réponse qui est proposé. Ensuite, la parole est à monsieur Bernard buis pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre l'attractivité des métiers de la fonction publique est un enjeu essentiel pour restaurer la confiance entre nos concitoyens et l'État. Le défi est de taille, notamment dans la fonction publique hospitalière. Pourtant des solutions existent, à l'image du développement de l'apprentissage à ce sujet. En ce qui concerne les agents de la fonction publique d'État, une prime d'apprentissage de 500 euros par an versés aux maîtres d'apprentissage a été créé par le décret du 27 septembre 2021. En ce qui concerne les agents de la fonction publique hospitalière de décrets ont été publiés le 9 et 20 septembre 2021 afin de rendre le dispositif d'apprentissage plus attractif, par le biais d'incitation financière des ces incitations sont dirigés vers les seuls établissements et il n'existe pas à ce jour de dispositifs individuels de valorisation des maîtres d'apprentissage. Or, de nombreuses collectivités territoriales à l'image du conseil départemental de la Drôme qui m'a alerté, ont décidé de s'engager dans la promotion de l'apprentissage afin de contribuer à une meilleure insertion professionnelle et de renforcer l'attractivité des métiers. Néanmoins, compte tenu de l'absence de dispositif individuels de valorisation des maîtres d'apprentissage au sein de la fonction publique hospitalière, certains employeurs ont actuellement recours à des méthodes inadaptées. Je pense notamment au paiement d'heures supplémentaires à destination des maîtres d'apprentissage ou encore à la prime de service. Il semble donc que les collectivités locales doivent traiter différemment les maîtres d'apprentissage de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État dans le ton texte difficile que traverse nos territoires en matière de couverture médicale crise en partie dû au manque d'attractivité des métiers de la fonction publique hospitalière. Il me semble donc important que le gouvernement puisse répondre sur ce sujet. Par conséquent, Madame la Ministre, quelles solutions pourraient être envisagées. Afin de mettre fin à cette discordance et ainsi dynamiser l'insertion professionnelle dans nos hôpitaux. Merci, cher collègue, la parole est à la ministre. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur. Bernard buis. Je vous remercie d'avoir bien voulu évoquer ce sujet important, le développement de l'apprentissage dans la fonction publique hospitalière est un enjeu clé participant activement à renforcer l'attractivité des carrières hospitalières, notamment vis-à-vis des jeunes pour qui cela représente une voie d'entrée privilégiée dans les carrières de la santé. La promotion de l'apprentissage au sein des établissements est nécessaire et constitue un levier bien identifiés par le gouvernement auquel il attache une importance prioritaire aussi pour répondre à l'objectif fixé de 4000 contrats d'apprentis dans la fonction publique hospitalière d'ici la fin du quinquennat. Une aide financière de l'État, d'un montant de 3000 euros par an et par apprenti sera mise en place pour le recrutement des apprentis dans la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, les services du ministère de la Santé et de la prévention mène actuellement des travaux afin de mettre en place sur le plan juridique, une allocation versée aux maîtres d'apprentissage au sein même de la fonction publique hospitalière, il était envisagé d'ouvrir le bénéfice de cette allocation d'ici la fin de l'année 2023. Madame la ministre, monsieur. Puis vous avez quelques secondes. Merci pour toutes ces précisions. Je pense que ça sera fortement apprécié. La parole est à présent à madame je suis guide. Pour sa question. Monsieur le président. Madame la ministre ma question se porte sur la réévaluation du pictogramme de femme enceinte annoncée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le 24 janvier dernier. Ce pictogramme est obligatoire sur toutes les boîtes de médicaments parmi lesquels la dépakine depuis 2017. Pendant des années, l'absence de signalétique a été trompeuse faisant croire aux patientes que le médicament était un produit comme les autres sans danger. Thalidomide distille ben dépakine les scandales liés aux médicaments sont nombreux et leur existence avait témoigné à de multiples reprises de la nécessité d'encadrer les pratiques et de prévenir des dangers pour qu'enfin ils cessent. Ce pictogramme vise ainsi à informer les femmes enceintes de la tératogène une cité d'un médicament et de limiter les risques pour leur enfant à naître. Celui-ci a notamment permis d'amener les femmes et dans un projet de grossesse à discuter des risques éventuels liés à la prise d'un traitement pendant la grossesse avec des professionnels de santé à réévaluer le traitement ou encore à se tourner vers une alternative thérapeutique en évitant les médicaments photo toxique. Il s'agit d'une information capitale pour anticiper et parfois même éviter aux femmes enceintes de recourir aux avortements médicaux. Or cette réévaluation n'intervient sans qu'aucune difficulté notable de compréhension n'ait été signalés par les patientes, madame la Ministre, pourriez-vous me préciser pourquoi. Et de quelle manière le conseil scientifique temporaire de l'ANSM en revue réviser ces pictogrammes clair simple à comprendre et utiles à la prévention des risques. Un retour en arrière n'est pas envisageable et risquerait d'entraver le consentement éclairé des patientes. Je souhaite aussi connaître la méthodologie de la révélation de ce dispositif ne serait-il pas plus pertinent de conserver en l'état les pictogrammes dans leur forme actuelle. Et si cette révélation sur la mise en place d'un observatoire ou d'un service dédié à leur opposition sur les bases sur les boîtes de médicaments, je vous remercie. De votre attention. Merci, cher collègue, la parole est à madame la ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice Guy Days vous m'interrogez sur la réévaluation du pictogramme de femme enceinte ce pictogramme représentant une femme enceinte barrée a été mise en place en 2017 et concerne les médicaments ou produits dont le résumé des caractéristiques cite des effets tératogène ou faites L'objectif recherché était de rendre les femmes enceintes vigilante et de les amener à se rapprocher de leur médecin ou pharmacien pour questionner la pertinence de la prise de traitement durant la grossesse et les accompagner dans l'évolution éventuelle de leur prise en charge. Cependant, des critiques ont pu émerger sur la bonne compréhension des visuels des retours de terrain ont notamment montré que certaines patientes pourraient pouvait arrêter brusquement leur traitement mettant leur santé en danger aussi l'ANSM a été saisi par la direction générale de la santé pour améliorer le dispositif et le rendre plus efficace dans l'intérêt des femmes. L'ANSM a mis en place un comité scientifique temporaire qui se réunit depuis janvier 2023. Son objectif est de faire un état des lieux de la compréhension de ce pictogramme par le public et de proposer un aménagement du dispositif réglementaire existant. Le comité réuni s'appuiera sur les les et les éléments suivants, pardon les résultats d'une enquête d'opinion diligentée par l'ANSM pour évaluer la connaissance et la réceptivité de ces pictogrammes les auditions les contributions écrites des différentes parties prenantes, les représentants des usagers professionnels consommateurs industriels et rédacteur de revues scientifiques à ce jour les auditions publiques de l'Apesac, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant du Conseil national de l'Ordre des Médecins de France assos Santé et des syndicats des industries pharmaceutiques ont été menées les prochaines auditions auront lieu fin mai 2023, à l'issue de ces travaux. L'évaluation de la faisabilité d'une évolution des pictogrammes sera évalué par l'ANSM et des propositions seront soumises au ministère pour validation avant leur mise en oeuvre, le cas échéant, une campagne de communication sera déployée par l'ANSM autour des pictogrammes revisité pour accompagner et améliorer l'appropriation du public. Merci madame la ministre. La parole est à présent la présidente Catherine Deroche pour sa question. Merci Merci monsieur le président. La loi Kouchner du 4 mars 2002 a rendu obligatoire l'assurance responsabilité civile des professionnels de santé, en prévoyant des plafonds de garantie. La loi à bout du. 30 décembre 2002. Opérer un changement de régime juridique substituant au principe dit base fait générateur. La garantie couvrant toutes les activités effectuées pendant la durée du contrat, celui de base réclamations plus de couverture indéfinie des actes de passer mais seulement d'effets dommageables non connu de l'assuré qui font l'objet d'une première réclamations par la victime pendant la période de validité du contrat en raison de trop de garantie pouvant résulter des dispositions. Combinées de ces de loi, l'article 146 de la loi de finances pour 2022 a créé un fonds de garantie de dommages consécutifs à des actes de prévention de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant un titre libéral c'est le F. Comme l'a constaté notre collègue Catherine Procaccia dans son rapport sur l'assurance. Responsabilité civile médicale de ces juin 2021 si la réforme conduite en 2012 avec la création de ce fonds et le relèvement des plafonds de garantie à 8 millions d'euros par sinistre a contribué à améliorer la couverture des professionnels de santé les plus exposés. Une question reste cette réforme a-t-elle mis fin à toute situation résiduel de toutes de trop de garantie pour des praticiens qui avait régulièrement souscrit une assurance responsabilité civile médicale. Ce sera le cas notamment de. De situations dans lequel la réclamation a été portée par la victime avant le 1er janvier 2012 ou en 2012 une enquête évalue à environ 5 médecins majoritairement des gynécologues obstétriciens, anesthésistes exposés à un risque de trop de garantie. Or la création permettait d'éviter de telles situations qui menace de ruine des praticiens concernés et leurs familles, je souhaiterais savoir ce que fait le gouvernement pour ces exclus. Merci madame la présidente, madame la ministre, votre réponse est attendue. Merci monsieur le président, madame, madame la sénatrice Catherine Deroche vous m'alerter sur les difficultés de médecins qui font face à des défauts de couverture assurantielle pour des montants individuels important et qui ne sont pas couverts par le F. PDS le fonds de garantie, abondé par les professionnels de santé. En effet le FA PDS intervient pour une réclamation soit déposée à compter du premier du 1er janvier 2012, en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance soit mettant en jeu un contrat d'assurance-conclut renouveler ou modifié à compter du 1er janvier 2012 en cas de dépassement des plafonds de garantie. Je suis sensible à la situation de ces médecins et de leurs familles néanmoins de par le nombre très limité de cas concernés que vous avez rappelé et conformément aux conclusions du rapport d'information de Madame. Catherine Procaccia 2002 1021 auquel vous faites référence, la situation n'appelle pas à ce jour une évolution des textes. Un élargissement des critères aurait en outre comme le souligne également le rapport de la sénatrice un impact non maîtrisée sur l'équilibre financier du Fonds et poserait un problème d'équité entre les professionnels qui cotisant au fond je souhaite toutefois que les travaux d'évaluation prospective soit relancée en lien avec les organismes concernés. Ces travaux de vont permettre de préciser la situation et le besoin de financement et d'ouvrir le cas échéant, une réflexion sur la mise en place d'un financement alternatif au FA PDS ou sur l'élargissement de certains critères de prise en charge. Si Madame la Ministre. La parole est à présent à madame Marie Mercier pour sa question. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre quel accueil voulons-nous pour nos petits-enfants dans les structures avant de vous parler du rapport de l'IGAS, je voudrais vous faire une remarque d'ordre général. Vous savez que les petits enfants arrivent dans les crèches quelquefois à 6h et demie le matin jusqu'à 11h 30, heure du déjeuner, ils ne peuvent rien manger et ceci même quand un pédiatre a pu diagnostiquer un retard c'est-à-dire au pondéral et réclamé cette alimentation du milieu de matinée. Vous en conviendrez c'est une aberration aberration absolue. Il y a d'autres façons de lutter contre l'obésité venons sont au rapport de l'IGAS du 11 avril il y a des dysfonctionnements graves, très graves dans certains établissements privation d'eau en font, qu'il ne faut pas changer. Nuisances sonores, aucune prise en compte du rythme du nourrisson. Ces enfants ont sont presque en danger. Pourquoi un constat aussi alarmant. Eh bien parce qu'il y a une logique comptable qui a prévalu sur le bien-être des enfants et que la pénurie de personnel et critique très critique. Avez-vous mesuré l'ampleur de cette crise, les professionnels de la petite enfance sont fois démotivés. Fatigués. Ils ont besoin d'être formés pour réagir aux difficultés et la qualité d'accueil des petits enfants dépend de l'équipe qui les prend en charge. La Fédération française des crèches a mis en avant aussi ses difficultés de recrutement, puisqu'y avoir des places fermées. Comment comptez-vous a accepté de fabriquer 200.000 places d'accueil alors qu'on manque de professionnels. Où en est le service unique de la petite enfance. Si cher collègue Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, madame la sénatrice Marie-merci. Je réponds bien volontiers à la demande de Jean-Christophe Combe, qui n'a pu être là ce matin en matière d'accueil du jeune enfant. Le précédent quinquennat a permis. Des avancées concrètes sur des sujets tels que la clarification des règles pour l'administration des médicaments, la création d'un référent santé accueil inclusive dans toutes les crèches ou la mise en place d'une charte obligatoire sur la qualité d'accueil. Le rapport de l'IGAS que vous évoquez que le ministre-Jean-Christophe Combe avait diligenté dès juillet dernier et qui l'a rendue publique il y a peu, nous invite néanmoins à aller plus loin. Il pointe notamment l'hétérogénéité de la qualité de l'accueil sur le territoire l'intégration insuffisante des connaissances sur le jeune enfant ou encore les limites des contrôles. Les propositions du rapport sont en cours d'expertise et le ministre s'est déjà engagé devant la représentation nationale ah y donner suite, dans les prochaines semaines. Sur ces questions. L'action du gouvernement est guidée par deux priorités, la première c'est de garantir à toutes les familles la meilleure qualité d'accueil dans tous les établissements publics, associatifs, privés en tenant compte des fragilités ou risque particulier identifié dans certains modèles. À ce titre, il n'est pas possible en raison de manque de personnel de respecter le cadre réglementaire. Il faut bien sûr réduire la capacité d'accueil et des décisions sont prises en ce sens par les préfets, suite notamment à la demande qui leur avait été faite dès l'été dernier par la Première ministre de se rapprocher des départements pour renforcer les contrôles, la 2ème priorité c'est de soutenir les équipes et de lutter contre la pénurie de professionnels à la fois le symptôme et facteur aggravant de la situation, le gouvernement, il travaille au travers d'une comité de filière dédiée avec une campagne de promotion des métiers et à la construction d'un socle social commun contrepartie de la participation de l'État au financement des revalorisations salariales. Ce que je résume là est en réalité c'est l'ambition de l'accueil de la garantie d'accueil du jeune enfant dont le ministre porte le déploiement, à la demande du président Laurent de la République et de la Première ministre et qui fera très prochainement l'objet de premières annonces. Si madame la ministre, Madame Mercier. Donc. Qui veut répondre. Bah, madame la Ministre, les crèches sont une chance pour le développement des enfants une chance absolue un État digne de ce nom. Ça doit être son honneur de protéger les plus vulnérables. Or, je vous remercie de vraiment porter cette petite histoire qui vous semble toute simple du côté de la matinée mais qui enfin fait partie de la santé de l'enfant. Merci de porter cela et de cette filière attractive. Merci, cher collègue, la parole enfin au président Guillaume Gontard. Merci monsieur le président, madame la ministre. Depuis plusieurs mois les hôpitaux isérois se trouve dans une situation alarmante à Voiron, un collectif de citoyens et de soignants cherche à interpeller le gouvernement sur le manque de moyens et de personnel. Alors que l'hôpital de Voiron et pratiquement 9 un bâtiment entier se retrouvent vide alors qu'il pourrait accueillir des lits pour prendre en charge les patients qui en ont besoin. Le CHU de Grenoble Alpes est également en grande difficulté. Les représentants du personnel en grève illimitée depuis plusieurs mois. Alerte sur leurs conditions de travail. Ils ont d'ailleurs déposé un signalement auprès de, auprès du procureur pour mise en danger de la santé d'autrui. Avec la fermeture des urgences de Voiron et de Bourgoin-je a lieu toutes les urgences du CHU de Grenoble Alpes sont complètement saturés. Conséquence dramatique de cette situation depuis décembre 2022, 3 personnes dont le pronostic médical indiquait pas d'urgence à leur arrivée sont décédés aux urgences en attente d'lit. L'équipe de chirurgie pédiatrique vient elle aussi de craquer nouveaux arrêts de travail oblige à annuler les interventions Piedra. Près de 500 enfants et leurs familles sont aujourd'hui dans l'attente, nous avons appris récemment que 123 lits seraient réouvert en septembre, mais cela ne compensera malheureusement pas le nombre de lits fermés, alors Madame la Ministre comptez-vous enfin prendre des mesures efficaces pour améliorer la situation du système hospitalier en France et notamment en Isère où elle est particulièrement critique. C'est pas évident. La parole est à la ministre pour cette dernière réponse. Merci monsieur le président, Monsieur le Sénateur, Guillaume Gontard, le gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures en réponse à votre question, pour améliorer la situation des systèmes de santé et des hôpitaux. L'investissement au Ségur la révélation des primes de nuit et des astreintes de garde notamment notre mobilisation est constante pour continuer de traduire les engagements du président en termes d'attractivité de refondation de nos hôpitaux au plan national comme au plan local. Certaines de ces mesures produisent déjà leurs effets, d'autres auront un impact à moyen terme la mise en oeuvre de ces mesures revient aussi aux acteurs territoriaux pour élaborer des solutions durables concernant la CHU, la situation du CHU de Grenoble Alpes les tensions existent principalement due à une pénurie de ressources humaines médicales et paramédicales plutôt qu'à un manque de moyens. Cependant, je ne peux pas vous laisser dire que la moitié des lits sont fermés. C'est faux. Et ces fermetures sont liés, tant à l'évolution des prises en charge qu'à des problématiques d'effectifs. Quant au signalement adressé au procureur, il a été classée sans suite. Je peux en revanche vous assurer que toutes les précautions sont prises par la gouvernance de l'établissement pour assurer la sécurité des patients en adaptant l'organisation aux ressources disponibles concernant le service des urgences du site de Voiron. Le service n'est pas fermé. Son organisation a été adapté sur les plages horaires de nuit du fait d'une insuffisance de ressources médicales concernant les locaux disponibles. Il ne s'agit pas d'un bâtiment entier vide mais d'une unité non utilisés en raison d'un projet initial d'installation d'une clinique voisine qui n'a pas été mené à terme ces espaces seront réaffectés à l'avenir en fonction des besoins de la population et des ressources disponibles. Le CH de Bourgoin reste opérationnel, offrant ainsi une solution alternative pour les patients. L'offre de soins urgents est également complétée par les cliniques privées dont les services d'urgences continuent de jouer leur rôle en réaction à ces tensions. Les mesures d'urgences, pérenniser issu de la mission flash sont pleinement mobilisés sur le territoire isérois. Celles-ci comprennent notamment l'envoi d'infirmiers à domicile par le SAMU pour les levées de doutes, la revalorisation des rémunérations pour encourager les praticiens à participer aux gardes et la régulation médicale entre autres ces actions appuyées par l'engagement des professionnels de santé permettent de garantir la continuité de la réponse aux besoins sur le de soins sur le territoire. Enfin, l'ARS joue un rôle dans la coordination des acteurs fluidifiant les filières de soins avec des avancées comme celles récemment obtenu dans la filière psychiatrique qui a permis de soulager le service d'urgences du CHU, Madame le ministre, et maintenant la parole pour finir est au président Gontard. que vous puissiez répondent de manière à la fois plus précises et surtout dans l'urgence actuelle parce que c'est maintenant et c'est toute de suite. Alors oui il y a une pénurie de ressources qui est liée notamment aux conditions de travail. On a beaucoup de médecins qui démissionne et avec un taux de postes vacants de 50 pour le CHU de Grenoble fonctionne aujourd'hui avec seulement la moitié des effectifs. Le problème n'est pas seulement financier, vous l'avez dit, les hôpitaux sont confrontés à des difficultés de recrutement il faut urgemment augmenter le nombre de places en année de Messine favoriser le recrutement extérieur en facilitant, par exemple, la reconnaissance de l'équivalence de formation des médecins étrangers. Merci. Merci cher président et. Merci madame la ministre je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 14h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casino. La séance est suspendue.